c'est avec une vive émotion que nous avons appris le décès du journaliste de l'Agence France-Presse (AFP) Arman Soldin, tué hier après-midi lors d'un bombardement dans l'est de l'Ukraine. Ce jeune homme de 32 ans risquait sa vie chaque jour au coeur du conflit pour nous informer. Au nom du Sénat tout entier, je présente nos condoléances à sa famille et à ses proches et je veux assurer de notre soutien l'ensemble des journalistes et techniciens qui exercent leur métier dans des circonstances particulièrement difficiles pour nous informer. aussi vive que nous avons appris l'attaque abjecte perpétrée à la synagogue de la Ghriba, à Djerba en Tunisie, qui a coûté la vie à quatre personnes, dont l'un de nos compatriotes, Benjamin Haddad.

je souhaite à mon tour, au nom du Gouvernement, exprimer toute mon émotion et ma solidarité après le décès, hier, en Ukraine, du journaliste Arman Soldin, qui couvrait le conflit pour l'AFP. Mes premières pensées vont à sa famille et à ses proches. Elles vont à ses collègues de l'Agence France-Presse. Elles vont à tous les journalistes. Arman Soldin accomplissait son métier, sa passion, sa vocation. Il est tombé parce qu'il voulait faire connaître des faits. Il est tombé parce qu'il croyait que le devoir d'informer ne doit reculer devant rien. Le journalisme, la presse libre sont essentiels pour nos concitoyens et notre démocratie.

Nous sommes donc face à une situation qui est loin d'être satisfaisante. Parallèlement, certains métiers ont du mal à recruter et ne trouvent plus de jeunes. La souveraineté industrielle, numérique et énergétique nécessite aussi de placer le lycée professionnel au centre de nos enjeux de formation et de repenser le parcours des lycéens. Le lycée professionnel doit donc redevenir, d'une part, un choix pour la plupart des jeunes à la recherche de métiers d'avenir et, d'autre part, une solution pour les entreprises qui doivent s'adapter aux grandes transitions économiques en cours et à venir. En faisant évoluer l'offre de formations proposée par les lycées, nous redonnerons du sens à la valeur travail et préparerons les compétences de demain, en adéquation bien sûr avec les aspirations des jeunes, de leur temps et du monde dans lequel ils vivent.

nous avons été choqués que vous ayez laissé se dérouler une manifestation non loin d'ici, en plein Paris, à la veille de la commémoration de la libération

Le racisme et l'antisémitisme n'ont pas leur place dans la République. Désormais, toute manifestation portant de tels messages sera interdite.

Il n'est certainement pas pertinent d'apporter la même aide à toutes les communes, quelles que soient leur taille et leur situation financière, mais la hausse du coût de l'énergie fragilise de très nombreuses collectivités. Il ne se passe pas une semaine sans que nous rencontrions des élus démunis face à des factures dont le montant a été multiplié par deux, trois ou quatre. Selon Intercommunalités de France, la facture d'énergie a au moins doublé pour les trois quarts des intercommunalités. Il y a sans doute une cote mal taillée qu'il serait bon d'ajuster, notamment pour les collectivités les plus en difficulté. La dotation globale de fonctionnement est repartie à la hausse après des années de gel ou de baisse, ce qui devrait donner un peu de marge aux élus locaux.

Je rappelle que les collectivités représentent 70 % de l'investissement public. L'enjeu est donc important. Il l'est d'autant plus que, pour réduire les factures d'énergie, l'opération de rénovation énergétique des bâtiments publics, déjà entamée, doit encore être accélérée,

Au 1 janvier de cette année, l'épargne brute de la totalité des collectivités locales avait progressé de 2,2 milliards d'euros par rapport au 1 janvier de l'année précédente, même si l'on constate des disparités entre les blocs de collectivités

près de 4 000 dossiers portent uniquement sur les questions de rénovation énergétique, auxquels il convient d'ajouter 2 500 dossiers concernant la rénovation de l'éclairage public. public. C'est dire si la volonté des élus de continuer d'investir et d'accélérer les rénovations énergétiques et thermiques est bien une réalité ! La Première ministre a annoncé la pérennisation de ce dispositif. Je recevrai le 17 mai toutes les associations d'élus,

Jeudi dernier, à Saintes, le Président de la République a présenté les détails de ce qu'il souhaite mettre en place : allongement de la durée des stages aux dépens des heures d'enseignements généraux, définition des formations par des « partenaires » et des entreprises, orientation des élèves vers les métiers en tension. Cela rejoint les propositions que vous portez depuis l'automne, madame la ministre. La concertation n'a pas fait évoluer les grandes lignes de la réforme. Seules nouveautés : des revalorisations inconditionnelles destinées à apaiser les enseignants mobilisés contre vos propositions

Beaucoup craignent aujourd'hui un rattachement pur et simple de la voie professionnelle au ministère du travail, ce qui constituerait une régression totale au regard de la mission émancipatrice du lycée.

Madame la ministre, nous sommes vraiment loin du programme des écologistes ! Vous proposez d'augmenter la durée des stages au détriment des enseignements généraux, ce qui revient, à nos yeux, à accroître les inégalités entre la voie générale et les voies professionnelles. Valoriser les stages en entreprise, c'est nier la force d'un enseignement associant formation générale et professionnelle. Adapter les formations aux bassins d'emploi, c'est renforcer les inégalités territoriales, en rendant les lycées dépendants du tissu économique local. Cette réforme mérite selon nous

Après avoir connu, ces dernières années, pendant deux ans, tous les samedis, les exactions des « gilets jaunes » - 140 manifestations en quatre ans ! -, les commerçants que j'ai rencontrés m'ont fait part de leur découragement, de leur peur et de leur colère. Certains, qui ont eu à subir plusieurs sinistres liés aux manifestations et aux casseurs, ont vu leur contrat d'assurance résilié. Ces commerçants retrouvent avec difficulté des compagnies d'assurances qui acceptent de les couvrir, ces dernières subordonnant le nouveau contrat à une période probatoire de deux ans sans sinistre. Ces commerçants n'ont plus qu'un seul choix, incroyable : celui de ne pas déclarer le dernier sinistre lié aux manifestations du 1 mai s'ils veulent conserver une couverture pour des risques plus graves dans la période probatoire imposée. Je sais combien Je sais combien cette situation préoccupe la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault et son président, qui, avec l'ensemble des commerçants, demande au Gouvernement de prendre des mesures législatives ou réglementaires afin de dissocier de toutes les autres clauses contractuelles les risques liés aux manifestations et aux casseurs. Ces commerçants demandent que soit garanti le maintien d'une couverture assurantielle dès lors que leur responsabilité ne peut être mise en cause. Ils sont les victimes de ces sinistres à répétition ; ils n'en sont pas les responsables.

ou de Paris pourraient décrire. Le Gouvernement déplore que les manifestations entraînent parfois des dégradations, mais également que ces difficultés emportent de lourdes conséquences pour les commerçants.

les dommages matériels, les assureurs sont en première ligne, les conséquences des dégradations étant prises en charge dans les contrats multirisques professionnels contractés par les commerçants. Quant à la garantie des pertes d'exploitation, elle peut être étendue aux conséquences d'autres événements que ceux qui sont prévus dans le contrat, comme les actes de vandalisme et les émeutes de manifestations, par exemple, à condition que ces événements soient intégrés au contrat. La couverture des dégradations liées à des manifestations n'est donc pas systématique. Nous estimons la part d'artisans et de commerçants couverts en cas de perte d'exploitation à 54 %. Plus les entreprises sont grandes, Concernant la résiliation unilatérale des contrats par les assureurs, la loi prévoit une telle possibilité en cas d'aggravation du risque, mais le Gouvernement veille à ce que des délais de carence d'incidents ne soient pas demandés aux commerçants.

J'ajoute que l'État est et restera également présent pour accompagner les commerçants touchés. Consigne a été donnée à la direction générale des finances publiques et aux Urssaf d'appliquer avec souplesse les modalités de remise gracieuse aux commerçants affectés par les manifestations et les dégradations.

le peuple ne supporte plus ces manifestations violentes. Aujourd'hui remonte du terrain un sentiment d'exaspération. Nous sommes en République, beaucoup l'ignorent.

À l'instar de milliers de familles des Alpes-Maritimes, j'ai été invité à étudier la proposition de l'inspection académique de permettre à mon fils de bénéficier de cours en arabe, en turc ou en portugais, dans le cadre des enseignements internationaux avec les pays dits « partenaires J'avais cru naïvement le Président de la République en 2020, qui avait dit lors de son discours sur le séparatisme à Mulhouse vouloir mettre fin aux dérives des enseignements de langue et de culture d'origine, les Elco. Or cette proposition de votre ministère, transmise aux familles, prouve que tel qui valide le choix des enseignants, de leurs qualifications, le contenu des enseignements, pour qu'ils soient respectueux de nos valeurs républicaines, alors que nous apprenons par la presse que les contrôles sont encore et toujours inopérants Pourquoi ne pas mettre fin aux risques de dérive communautariste, comme le pointaient déjà nos collègues sénateurs dès 2003 ? Pourquoi, tout simplement, ne pas en finir avec les influences étrangères ? Ces enseignements clivent au lieu de rassembler et, surtout, encouragent le repli communautaire. Monsieur le ministre, prenons-nous véritablement le bon chemin de l'intégration en dispensant aux élèves des écoles primaires l'arabe, ou encore le turc, langue d'un pays avec lequel nous ne partageons aucune frontière, peu de valeurs, et dont l'influence en France est inquiétante ? Alors que le niveau de nos élèves est en constante diminution, ne serait-il pas préférable de nous recentrer sur l'accès aux savoirs fondamentaux et sur une seule et véritable priorité, à savoir la maîtrise de la langue française ?

et le discours du Président de la République sur le séparatisme à Mulhouse, les enseignements internationaux de langues étrangères ont remplacé les enseignements de langues et de cultures d'origine.

Non, pas l'italien ! Afin d'éviter toute dérive communautaire ou toute influence étrangère, ce nouveau dispositif a permis d'instaurer un cadre homogène fondé sur un accord bilatéral entre les pays. Il a également permis d'imposer que les enseignants aient un niveau minimal de langue française, contrôlé dès leur entrée en fonction à un niveau B2

plutôt que dans d'autres lieux, qui ne seraient pas nécessairement adéquats. Cet enseignement, qui concerne environ 70 000 élèves, soit à peu près 1 % des enfants de l'école élémentaire, se déroule désormais dans des conditions acceptables.

Pourtant, j'ai toujours été fier de dire que j'avais fait mon cursus scolaire au sein de l'école publique. J'avais le même souhait pour mes enfants, mais vous contribuez fortement, malgré des enseignants méritants, à faire de notre école un lieu de séparatisme, de communautarisme et d'échec scolaire

Ma question porte sur les craintes des maires concernant de nouvelles vagues de fermetures de bureaux de poste dans les communes rurales, mais aussi dans les communes

souhaité conforter la présence postale dans un contexte- vous l'avez souligné -de baisse significative de la fréquentation des guichets, en accompagnant notamment le déploiement du dispositif France Services, sur lequel veille

accompagner le développement des usages numériques et de la médiation sociale à destination des populations les plus vulnérables. Enfin, nous avons souhaité optimiser les règles de gouvernance et de fonctionnement des commissions départementales, pour une meilleure utilisation du fonds de péréquation. J'ajoute que les actions qui figurent dans ce contrat doivent bénéficier de manière prioritaire aux zones rurales, aux zones de montagne, aux quartiers prioritaires de la politique de la ville et aux outre-mer. Par ailleurs, l'État a indiqué son intention de poursuivre son soutien, en complément des abattements fiscaux, au moyen d'une dotation budgétaire dont le montant sera déterminé dans le cadre des projets de loi de finances pour 2024 et pour 2025. Nous aurons donc l'occasion d'en débattre ici. Vous le voyez, monsieur le sénateur, le Gouvernement veille à ce que la présence postale sur les territoires reste intacte. Monsieur le ministre, vos propos sont implacables, mais il est essentiel dans ce domaine de ne pas pécher par excès de rationalité. Le service postal dans notre pays est un symbole de l'État et de sa présence territoriale.

Ma question s'adressait à M. le ministre délégué chargé des comptes publics, mais je sais qu'il est empêché et que c'est M. le ministre Lescure, chargé de l'industrie, qui me répondra. Le ministre Attal fut hier dans tous les médias afin de présenter son plan de lutte contre la fraude fiscale. Il a déclaré vouloir « faire faire payer les impôts aux ultra-riches et aux multinationales qui fraudent ». Fichtre, voilà un discours auquel nous n'avions pas été habitués depuis 2017 ! Vous étiez, en effet, plutôt sur le registre de. Vous Vous annoncez vouloir renforcer le service d'enquête judiciaire, mais dans le même temps la direction générale des finances publiques va subir 3 000 suppressions d'emplois supplémentaires d'ici à 2027. Nous notons avec intérêt l'idée d'une COP de la fiscalité et la création d'un conseil d'évaluation, sans doute une nouvelle mouture de l'observatoire imaginé par votre illustre prédécesseur en septembre 2018, une instance qui n'a malheureusement jamais vu le jour. Je crains, monsieur le ministre, qu'il n'y ait un angle mort majeur dans votre dispositif : les paradis fiscaux. Considérez-vous, comme Bruxelles, qu'il n'existe pas de paradis fiscal au sein de l'Union européenne Souvenez-vous un peu des révélations du journal en février 2021 dans l'affaire OpenLux. Nous y apprenions que le Luxembourg hébergeait 55 000 sociétés offshore, dont 17 000 détenues par des compatriotes français cumulant ensemble 6 500 milliards d'euros d'actifs. On ne peut pas, à cet instant, évoquer la fraude fiscale sans parler d'évasion fiscale. Allez-vous prendre des initiatives à l'échelon européen sur ce sujet ? N'y a-t-il pas lieu de mettre sérieusement à jour la liste française des paradis fiscaux, qui comprend aujourd'hui des États aussi fondamentaux- n'y voyez aucune marque de mépris de ma part -que le Vanuatu, les Palaos et les Fidji,

je n'ai pu m'empêcher de sourire en imaginant un instant le PDG d'Amazon, M. Jeff Bezos, un pinceau à la main, en train de repeindre les murs de la perception d'Armentières, dans le Nord, dans le cadre d'une peine de travaux d'intérêt général

les relations et le travail de coopération à l'échelon international pour traquer la fraude fiscale là où elle se trouve. Depuis six ans, le Gouvernement a fait des choses sur ce sujet. Lesquelles ? Si les multinationales sont désormais taxées à un niveau minimal

Elle indique également les étapes à suivre pour pouvoir évaluer cette trajectoire. Surtout, elle précise que, en concertation avec les parties prenantes, notamment les collectivités, le Gouvernement peut définir et de la maîtrise de l'énergie (Ademe), prévu et attendu en 2023, et après évaluation des impacts environnementaux et économiques, les modalités d'une éventuelle mise en oeuvre de la consigne. Tel était le préalable indispensable à toute décision sur la consigne, que l'on y soit favorable ou non.

Les parties prenantes, particulièrement les élus, s'inquiètent et s'interrogent, surtout au regard des investissements lourds engagés dans leur territoire en faveur de la transition écologique. Ma question, monsieur le ministre, est simple : quelles sont franchement vos intentions ?

La région Île-de-France et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par exemple, sont aux alentours de 40 % pour les bouteilles en plastique contre une moyenne de 60 %. À l'inverse, la Bretagne et les Pays de la Loire sont à plus de 70 %. Un département comme la Haute-Saône a même déjà atteint 90 % de recyclage des bouteilles en plastique. C'est dire si, dans ce domaine, nous devons aussi nous inspirer de ce qui fonctionne ! La concertation vise, à la fois, dans le cadre de groupes de travail nationaux, à examiner comment faire plus et mieux

La parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, l'inflation s'est installée durablement à un haut niveau dans notre société. De très nombreux Français vivent au quotidien une austérité de fait, qui affecte sensiblement leur pouvoir de vivre. Alors que les défis environnementaux et sociaux sont immenses, le rétablissement des comptes publics ne doit pas se faire au détriment de l'action publique, celle de l'État comme celle des collectivités, qui sont en première ligne auprès de nos concitoyens. Au terme de l'année 2023, l'inflation se sera traduite par une perte, en euros constants, de plus de 1 milliard pour la seule L'inflation est très supérieure à 10 % pour le panier du maire, et elle va durer. À ce niveau, vous ne pouvez pas laisser l'action publique locale s'affaiblir durablement. Dans ce contexte, les élus constatent que les filets de sécurité et autres amortisseurs ont des limites. En matière d'investissement, des préfectures enregistrent des taux de réalisation d'à peine 60 % sur le cycle de mandat et rendent des crédits. Il n'est pas normal que des collectivités renoncent à l'action pour cause de capacité d'autofinancement dégradée par la conjoncture ou de complexité administrative de gestion des dossiers.

Madame la ministre, quelles mesures structurelles et durables envisagez-vous de prendre pour préserver, voire pour restaurer, les capacités de fonctionnement et d'investissement de nos collectivités locales ?

pour la première fois depuis treize ans, et vous le savez bien, le Gouvernement a décidé d'une hausse exceptionnelle de 320 millions d'euros en loi de finances, qui a permis à 90 % des communes de voir leur DGF augmenter. Dans la ruralité, que vous connaissez bien,

! Ces hausses de DGF s'ajoutent à l'ensemble des mesures décidées en loi de finances pour 2023 pour soutenir les finances des collectivités territoriales. Je pense au bouclier tarifaire, à l'amortisseur électricité, au filet de sécurité, au maintien des dotations d'investissement à leur plus haut niveau, à la création du fonds vert et à la revalorisation des bases de fiscalité locale à hauteur de 7 %. que, pour 2023, la somme des mesures prévues pour les collectivités a été plus importante qu'une simple indexation de la DGF sur l'inflation : 2,8 milliards d'euros ont été inscrits en loi de finances initiale pour 2023 alors qu'une indexation sur la DGF n'aurait conduit qu'à une augmentation de 1,1 milliard d'euros en 2023. Cet effort significatif témoigne de la volonté du Gouvernement d'apporter un soutien continu aux communes, particulièrement à celles qui sont confrontées à des difficultés économiques et sociales. L'intégralité des conséquences de l'inflation doit faire l'objet d'un effort commun des collectivités territoriales

pour ma part, qu'elles seront partie intégrante du plan d'austérité que vous êtes en train de mettre en place. À l'inverse, nous pensons que, pour répondre aux besoins des Français, les moyens des collectivités doivent être préservés à tout prix. Avec les élus locaux, nous restons dans l'attente de mesures rapidement efficaces.

pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Monsieur le ministre, 430 000 élèves sont reconnus en situation de handicap, soit en moyenne un élève par classe. Il est de la responsabilité de votre ministère, mais c'est aussi une question de justice sociale, d'humanité et d'honneur pour notre pays, d'accompagner au mieux ces enfants et adolescents vers plus d'autonomie et vers la réussite scolaire.

Toutefois, en l'absence d'une organisation adaptée et d'une véritable approche éducative centrée sur les besoins spécifiques de ces élèves, notre système a atteint ses limites et ne permet pas de répondre aux attentes des enfants et des familles concernés. Il met même parfois l'institution scolaire en difficulté. Dans un récent rapport que j'ai rendu au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat, nous appelons à franchir une nouvelle étape dans la mise en oeuvre d'une politique d'inclusion scolaire efficace formulons une vingtaine de préconisations. Nous vous proposons de mettre en place un cadre culturel rénové et une organisation administrative profondément corrigée, en faisant de l'accessibilité pédagogique la priorité qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, en prônant une prise en charge des élèves plus qualitative et continue, en améliorant les relations avec les familles, en renforçant les liens avec le secteur médico-social, ainsi qu'en respectant et en professionnalisant le beau métier d'AESH. Alors que la Conférence nationale du handicap a créé plus de déceptions qu'elle ne suscite d'espoir, monsieur le ministre, êtes-vous prêt à travailler sur la base des propositions du Sénat à à la création d'un véritable service public de l'inclusion scolaire

qui s'est tenue le 26 avril dernier, propositions très substantielles -nous aurons l'occasion d'échanger ensemble à ce sujet. Dès la rentrée 2023, tous les enfants scolarisés, y compris ceux qui

Nous avançons du côté du périscolaire avec les collectivités, mais nous proposons aussi de rapprocher les AESH de la vie scolaire et des assistants d'éducation de manière à augmenter leur temps de travail, à les attacher à un établissement et à enrichir leur métier.

Union Centriste. Ma question s'adresse à M. le ministre de la santé et de la prévention. Dynamiques tout au long de la crise sanitaire, les collectivités ont demandé à participer plus activement à la gouvernance des agences régionales de santé (ARS) pour mieux coordonner les réponses institutionnelles sur le terrain.

Cette mesure vise à renforcer l'ancrage territorial de ces établissements publics, ainsi que le rôle des parlementaires, afin de corriger le fonctionnement d'une administration trop centralisée. En tant que membre du Sénat, j'ai été désignée le 22 avril 2022 par le président Gérard Larcher pour siéger, avec voix consultative, au sein du conseil d'administration de l'ARS Île-de-France. Ma collègue Nadia Sollogoub, que j'associe à ma question, l'a été pour l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. N'ayant pas reçu de convocation, à l'instar de tous mes collègues sénateurs, pour participer aux réunions de cette instance, j'ai découvert à ma grande surprise que les décrets d'application organisant l'évolution de ce conseil n'ont pas été publiés à ce jour. Par conséquent, la direction des ARS ne peut pas modifier le fonctionnement actuel. Pour contribuer aux projets qui répondent aux besoins des territoires, notamment pour faire face au défi de la désertification médicale, les membres titulaires de ce futur conseil d'administration attendent impatiemment la publication de ces décrets. Pourriez-vous, monsieur le ministre, m'apporter plus de précisions à ce sujet et m'indiquer votre plan d'action pour accélérer l'évolution de ces dispositions ? La parole est à M. le ministre de la santé et de la prévention. Madame la

et de la cohésion des territoires, le 15 avril dernier, la Caisse des dépôts et consignations, propriétaire de nombreuses forêts, a suspendu tous ses chantiers jusqu'à nouvel ordre. La direction interdépartementale des routes, qui veille à la sûreté routière, Ces arrêts font suite à une décision de l'Office français de la biodiversité (OFB), qui se fonde sur l'article L. 411-1 du code de l'environnement, lequel permet d'interdire toute destruction d'habitat et de suspendre tout chantier en forêt ou sur bosquet.

Ces entreprises nous alertent, car elles se retrouvent sans activité pendant une période minimum de cinq mois, non définie, et dépendante de l'arbitrage de l'OFB. dorénavant incapables d'exploiter les bois en milieu humide, de réaliser en sept mois les travaux annuels et de produire le besoin national en bois. Dois-je vous rappeler, monsieur le ministre, que les entreprises du bois contribuent à la protection contre les incendies, comme nous l'avons souhaité dans le texte visant à renforcer la que nous avons connus en 2022 ? Le bois est aussi le matériau nécessaire à la construction et à la lutte contre la précarité énergétique des logements. La pénurie créera de l'inflation et contribuera à la crise du logement naissante. Enfin, le bois est une source d'énergie renouvelable nous permettant de lutter contre la dépendance aux énergies fossiles. Sans exploitation temporaire, les entreprises vont devoir recourir au chômage partiel, arrêter leurs investissements, voire se mettre en cessation d'activité. Seront-elles les prochaines victimes de la désindustrialisation de la France ? De plus, l'interprétation de l'article du code de l'environnement par l'OFB, qui voit un danger dans tout chantier en forêt, me paraît abusive et éloignée de la volonté du législateur. législateur. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire dans un futur immédiat et de façon durable pour les entreprises du bois qui, comme toutes les autres, ne peuvent vivre sans travailler ? La parole est à M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

à la fois un moyen de réindustrialisation, de soutien à la décarbonation et de stockage de carbone. Cette brique essentielle de la planification écologique a été précisée, sous l'autorité de la Première ministre.

forêt-bois de réunir l'ensemble des acteurs concernés- les ONG et toutes les entreprises sylvicoles -, en liaison étroite avec le ministère de l'agriculture, compétent s'agissant de la récolte sylvicole.

et Républicain. Ma question s'adresse à M. le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Après des années d'immobilisme gouvernemental lors du quinquennat précédent, il aura fallu un drame pour que vous vous saisissiez du sujet de la petite enfance et des crèches.

à la fois la maltraitance institutionnelle qui pèse sur les professionnels, un taux d'encadrement trop faible, une formation insuffisante des personnels, des modes de financement inadéquats, une gouvernance et un contrôle qui doivent être renforcés.

ce qui a conduit, ces dernières années, à « une dégradation progressive de la qualité d'accueil au profit de logiques financières ». Après les hôpitaux, les Ehpad, c'est au tour des crèches d'être délaissées par la puissance publique, et ce au profit de la logique marchande. Monsieur le ministre, quand allez-vous enfin reformer le secteur de la petite enfance et investir pour permettre à chaque enfant d'être accueilli dans des conditions qui garantissent son développement et son bien-être ?

vous avez raison, la sécurité des enfants accueillis doit être la première de nos priorités collectives. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dès que j'ai été nommé ministre, en juillet dernier, j'ai diligenté une mission de l'inspection générale des affaires sociales pour faire la lumière sur la situation dans les crèches et nous assurer de la robustesse des règles qui y sont appliquées, ainsi que de la qualité des contrôles. J'ai également demandé que les inspecteurs nous fassent un certain nombre de propositions.

mais aussi au manque d'intégration des connaissances sur le jeune enfant dans les projets d'établissement et dans la formation des professionnels. Enfin, le rapport met au jour les limites des contrôles qui sont assurés aujourd'hui

pas d'intentions vagues et sans calendrier. Il faut conclure ! Il est temps de mettre en place un véritable service public de la petite enfance. La parole est à M. Christophe-André Frassa, pour le groupe Les Républicains.

pour de prétendues atteintes à la sécurité intérieure de l'État, pour complot et espionnage. Notre compatriote a été maintenu dans un premier temps en détention provisoire, ce qui a légitimement provoqué des tensions entre la France et la République

Juan Rémy Quignolot a entamé une grève de la faim pour dénoncer sa situation. Les allégations fantaisistes portées contre lui ne peuvent en aucun cas constituer le fondement d'une enquête judiciaire sérieuse.

d'une relation délétère entre la France et la Centrafrique. Rien de plus ! Nous ne pouvons pas l'accepter ! Ce triste anniversaire doit être le dernier et la France doit tout mettre en oeuvre pour que Juan Rémy Quignolot retrouve sa liberté et son pays.

de sa mise en liberté provisoire, afin qu'il puisse recevoir les soins médicaux nécessaires dans l'attente de son procès. Ce que je peux vous dire, c'est que, durant sa détention provisoire, M. Quignolot a bénéficié de ce que l'on appelle la protection consulaire, prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963. Il a reçu, à ce titre, un certain nombre de visites consulaires. Sa situation continue d'être suivie quotidiennement à la fois à Bangui et à Paris, et les services du Quai d'Orsay sont en relation étroite avec sa famille. Ils suivent la situation et nous espérons évidemment une résolution rapide de son cas.

provenant de la France entière convergent vers un terrain privé de l'association Vie et Lumière. En 2022, ils étaient plus de 30 000 et, depuis le 6 mai dernier, ils sont plus de 40 000 voyageurs dans une commune de 1 200 habitants, au sein d'un bassin de vie de 25 000 personnes autour de la petite ville de Gien. Faute de places, des gens du voyage occupent illégalement des terrains agricoles, branchent leurs installations électriques et d'eau directement chez des particuliers, et les alentours, devenus un véritable cloaque, sont jonchés d'immondices en tout genre. De fortes tensions sont en train d'éclater entre les habitants excédés et des gens du voyage. Cette situation pose de graves problèmes de sécurité, de salubrité et de santé publiques, d'autant que les urgences de l'hôpital de Gien sont fermées jusqu'au mois de septembre prochain, faute de personnel. Aucun des services publics n'est dimensionné pour un tel afflux. Jusqu'à présent, les élus acceptaient le principe d'un unique rassemblement, dès lors que celui-ci respectait les capacités du terrain, soit 20 000 personnes. Ce n'est plus le cas et, depuis quelques années, un second rassemblement de gens du voyage venant de toute En 2015, les élus locaux et les parlementaires, dont nos collègues Sueur et Cardoux, avaient déjà alerté le Premier ministre, lequel s'était engagé à ce que l'État propose dorénavant un autre lieu pour un second rassemblement annuel. La promesse fut respectée pendant quelques années, mais elle ne tint qu'un temps. Depuis, les élus ont été promenés dans différents ministères et ont été reçus par plusieurs premiers ministres. En vain ! L'ensemble des habitants subissent au quotidien, nuisances et incivilités, et la commune de Nevoy demeure isolée. Madame la ministre, pouvez-vous en priorité faire respecter la parole de l'État ? Comptez-vous faire preuve d'autorité pour enfin enfin reprendre le contrôle de cette situation inadmissible

Ce rassemblement évangélique, qui se déroule cette année du 6 au 14 mai, devait accueillir environ 20 000 personnes. Elles sont aujourd'hui plus de 40 000, comme vous l'avez indiqué, dans une commune de 1 200 habitants. Cela fait peser sur cette dernière et les services de l'État une très forte contrainte. Je tiens à saluer l'implication des élus et des services de l'État pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions.

perspective d'un second rassemblement au mois d'août. J'entends les inquiétudes des riverains et des élus. Je le répète, le Gouvernement est pleinement mobilisé sur ce sujet. Je m'engage à ce que l'ensemble des parties prenantes- élus, associations d'élus, association Vie et Lumière -soient associées pour dégager des solutions pour les années à venir, dans le respect des sensibilités de chacun. La parole Le Gouvernement fuit ses responsabilités, abandonne et livre à eux-mêmes les habitants de Nevoy. Ainsi, vous actez la totale démission de l'État pour protéger ses citoyens.

La séance est reprise. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande de la commission des finances tendant à obtenir du Sénat, en application de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qu'il lui confère, pour une durée de trois mois, les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener une mission d'information portant sur la création du fonds Marianne, la sélection des projets et l'attribution des subventions, le contrôle de leur exécution et les résultats obtenus au regard des objectifs du fonds. Il a été donné connaissance de cette demande au Sénat lors de la séance du 3 mai dernier.

les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête pour mener cette mission d'information. Le Gouvernement sera informé de la décision qui vient d'être prise par le Sénat. L'ordre du jour appelle les explications de vote et le vote sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer (projet n° 540, texte

Toutefois, dans un souci de simplification et d'intelligibilité des règles juridiques, nous avons finalement préféré une nouvelle présentation et une réécriture de la quasi-totalité des articles.

dispositions du projet de loi sont applicables de plein droit aux départements, régions et collectivités ultramarines relevant de l'article 73 de la Constitution- la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte -, régies par le principe d'identité législative,

Pour les collectivités du Pacifique, soumises au principe de spécialité législative, relevant de l'article 74 de la Constitution- la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna -et pour la Nouvelle-Calédonie, les lois et règlements n'y sont applicables que dans les matières relevant statutairement de la compétence de l'État et sur mention expresse. Or c'est le cas en matière bancaire et financière. Les dispositions du projet de loi y sont donc applicables, sur mention expresse.

du 15 février 2022, qui a été prise sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution, prévoit une habilitation permanente pour étendre à l'outre-mer les dispositions législatives déjà existantes qui ressortent de la compétence de l'État,

et qui porte diverses dispositions relatives à l'outre-mer, vous est soumis après son examen attentif par la commission des finances. Une fois adopté, il permettra d'achever la refonte du livre VII du code monétaire et financier.

devenu illisible au fil des évolutions apportées par le législateur et par la transposition du droit de l'Union européenne. L'une de ces ordonnances a été prise sur le fondement de l'habilitation permanente, prévue à l'article 74-1 de la Constitution, lequel prévoit que les ordonnances prises sur son fondement deviennent caduques en l'absence de ratification par le Parlement dans un délai de dix-huit mois suivant leur publication. Voilà pourquoi la ratification de ces deux ordonnances nous est proposée aujourd'hui.

les modifications de certains articles du code monétaire et financier intervenues après la publication des ordonnances. Sur ce point, la commission s'est contentée d'adopter un amendement rédactionnel.

qui met en oeuvre la politique monétaire dans la zone du franc Pacifique. Les articles 7 et 8, qui apportent des modifications d'ampleur modeste aux missions de ces deux instituts,

et au suivi des comptes détenus par les personnes physiques et morales sur lesquels peuvent être tirés des chèques. Il est prévu dans les articles 7 et 8 que le Ficom soit élargi aux comptes de toute nature et aux locations de coffres-forts. La commission des finances a adopté l'amendement de suppression de l'article 9 proposé par M. le rapporteur, et ce pour trois raisons.

Deuxièmement, le Ficom a déjà une existence législative, qui est renforcée dans le cadre du présent projet de loi. Troisièmement, l'encadrement des modalités d'accès n'était pas conforme à celui qui était prévu pour le Ficoba ou pour

qui procèdent à diverses corrections, ainsi que des articles 10 et 11, le premier mettant à jour la numérotation des articles, le second différant l'entrée en vigueur de plusieurs dispositions.

le présent projet de loi, examiné selon la procédure de législation en commission, ne fait pas partie de ces textes qui déchaînent les passions. Il ne donnera pas lieu à de grands affrontements politiques. Sa technicité nous oblige à la plus grande modestie. Certains, à l'image de M. le rapporteur, ont déploré des délais d'examen réduits, mais la commission a salué le travail de fond et de réécriture. Les délais permettent au Gouvernement de demander la ratification du texte dans le délai imparti par la Constitution. Ce texte répond avant tout à une obligation constitutionnelle de ratification de trois ordonnances. Ce sont autant d'ordonnances qui ont permis de simplifier, de corriger et de regrouper des articles de loi souvent épars

le plus difficile pour le législateur est de garder une vision d'ensemble de notre droit, afin qu'il reste simple et lisible, alors même qu'il est traversé par nombre de notions complexes et de principes parfois contradictoires. Ce droit est avant tout un outil pratique pour l'administration, pour le juge, pour l'auxiliaire de justice et pour le justiciable. Ils doivent être en mesure de le connaître et de le comprendre pour pouvoir s'y conformer. Trois années d'un long et fastidieux travail ont été nécessaires pour parvenir à simplifier et à corriger un droit financier souvent trop complexe.

Je ne m'appesantirai pas sur la prolongation de l'expérimentation introduite par M. le rapporteur visant à permettre aux collectivités de recourir au financement participatif

de cohérence légistique, ne posent pas de difficultés majeures. Tout ce travail de codification, que nous nous apprêtons à avaliser aujourd'hui, permettra, à mon sens, de rendre plus accessible notre droit, qui s'est considérablement complexifié, sous l'effet des crises financières majeures, telles que celle de 2008. Tout ce travail de simplification facilitera surtout- c'est bien là l'essentiel -l'activité des opérateurs financiers et des entreprises outre-mer. Ainsi, j'espère que les corrections auxquelles nous avons permettront d'interroger utilement le Parlement et le Gouvernement sur l'intelligibilité et l'efficacité des lois que nous construisons pour nos concitoyens.

Au-delà de ces considérations, je me permets de mettre un bémol à ce satisfecit global. Je regrette, en effet, que nous adoptions l'article 5 relatif à la tarification des retraits d'espèces dans un distributeur automatique.

Concertation et célérité ne sont pas antinomiques. Nous souhaitons donc que le Gouvernement améliore son action dans les outre-mer. Pour autant, nous voterons ce texte. La parole est à M. Éric Bocquet, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste. madame la ministre,

fustigeant des saisines multiples et en urgence. Elle a été contrainte d'émettre un avis défavorable sur ce texte, car « la méthodologie employée par l'État continue de nuire gravement à l'intelligibilité du droit en matière monétaire et financière, car elle rend impossible, faute de temps et de concertation, d'évaluer les effets des modifications proposées ».

s'agit de permettre aux collectivités d'émettre des obligations à des créanciers qui pourraient être des personnes morales, donc des entreprises. Cela revient à faire financer tous les services publics choisis par les collectivités par les entreprises une plateforme en ligne.

L'affectation budgétaire des montants collectés est interdite, car elle entre en contradiction avec le principe d'universalité budgétaire. La promesse politique d'utiliser cet argent pour un investissement particulier est possible, mais elle n'est soumise à aucune contrainte juridique. L'universalité budgétaire est la manifestation d'une solidarité. Total finançait les services publics de la petite enfance ou les services environnementaux. À l'avenir, Total pourrait choisir de financer un service public selon ses propres intérêts. Il en va de même pour les impôts locaux aux personnes physiques

Donner cette responsabilité aux entreprises, c'est mettre en concurrence le système bancaire avec des entreprises, qui tiendraient en joue les finances locales. À terme, il en résulterait un désengagement budgétaire de l'État.

ailleurs, l'article 5 vise à revenir sur la gratuité des opérations de retrait d'espèces en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Le Gouvernement évoque un recentrage dans l'étude d'impact, tandis que Bercy parle, en, d'une erreur. Que disent les assemblées concernées, si ce n'est qu'elles n'y sont pas opposées ? C'est un signal négatif envoyé aux habitantes et aux habitants de ces territoires, qui auraient pu constater une avancée- une seule ! -, dans un contexte de diminution du nombre de distributeurs de 8,7 % entre 2018 et 2021 en métropole,

Ces frais, qui comprennent les frais de tenue de compte, l'abonnement à la consultation des comptes, les frais de paiement et les cartes à débit immédiat restent tout de même deux fois plus élevés là-bas qu'ici en métropole ou qu'en Nouvelle-Calédonie. Le maintien de la gratuité des opérations de retrait aurait de ce fait été un moyen de compenser l'asymétrie

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous sommes amenés, cet après-midi, à nous prononcer en première lecture sur le projet de loi ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer, examiné suivant la procédure de législation en commission prévue par notre règlement. Le recours à cette procédure s'est avéré une fois de plus fructueux, et je tiens à saluer la qualité du travail de notre rapporteur, dont il faut bien avouer que la tâche n'a pas été facilitée par le Gouvernement. En tant que parlementaires, nous ne pouvons pas nous satisfaire d'un délai d'examen aussi bref, à plus forte raison lorsque celui-ci empiète sur la suspension de nos travaux. Nous nous permettons d'insister sur ce point, car ce n'est pas la première fois que le travail du Parlement se trouve ainsi entravé. Vous en conviendrez, madame la ministre, là n'est pas le meilleur moyen d'assurer le bon fonctionnement de la démocratie représentative ni d'impliquer et de respecter les collectivités concernées. J'en viens au fond du texte, essentiellement technique, mais assez touffu, et dont la plupart des dispositions ne soulèvent pas de difficultés particulières. Je ne reviendrai pas sur les articles 3 à 8 ni même sur les articles 10 et 11, qui, procédant à des corrections purement formelles ou à des modifications extrêmement limitées, n'appellent pas de commentaires particuliers. Les articles 1 et 2 sont, en revanche, plus substantiels. L'article 1- cela a été rappelé par les orateurs précédents -procède à la ratification de trois ordonnances. Les deux premières, en date respectivement du 15 septembre 2021 et du 15 février 2022, sont prises sur la base d'une habilitation qu'avait soutenue le Sénat lors de l'adoption de la loi Elles permettent d'organiser de façon thématique le livre VII du code monétaire et financier, devenu abscons à la suite des modifications apportées par le droit national et par le droit européen. Le contenu de l'ordonnance a été scindé en deux par le Gouvernement afin de respecter le délai d'habilitation octroyé par le Parlement. Ce travail de recodification fut, certes, long et fastidieux, mais il se révèle utile, en ce qu'il offre aujourd'hui davantage de clarté et une meilleure lisibilité au droit applicable aux collectivités du Pacifique. Je partage toutefois les interrogations du rapporteur sur la méthode retenue par le Gouvernement. Nous ne pouvons que nous associer aux critiques émises par Moihara Tupana et par notre collègue Teva Rohfritsch, tous deux membres de l'Assemblée de la Polynésie française, s'agissant des saisines rectificatives multiples faites par l'exécutif dans la précipitation. Là encore, la forme trahit une impréparation du Gouvernement qui soulève quelques interrogations. La troisième et dernière ordonnance ratifiée par l'article 1, en date du 14 septembre 2022, a trait au financement participatif. Il est ici question de prolonger le délai de transition laissé à l'ensemble des acteurs du secteur, au-delà donc des seules collectivités ultramarines. Saluons la prolongation de deux ans, sur l'initiative du rapporteur, de l'expérimentation visant à ouvrir le financement participatif obligataire aux collectivités territoriales. En garantissant une expérimentation effective de trois ans, l'amendement adopté en commission permet, du même coup, de respecter la volonté du Parlement exprimée en 2021 dans le cadre du projet de loi portant Enfin, je me contenterai de mentionner l'article 2, bienvenu lui aussi, puisqu'il rend expressément applicables aux collectivités du Pacifique les modifications de certains articles du code monétaire et financier intervenues postérieurement à la publication des ordonnances.

Sans surprise, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les membres du groupe Union Centriste voteront les dispositions de ce texte tel qu'il a été amendé et adopté en commission, sur proposition notamment de notre ami et rapporteur Hervé Maurey. La parole

Si une banque suspecte un client de malversations, il est normal qu'elle alerte les services fiscaux ou la justice. En revanche, ce n'est pas à elle de conduire une enquête et encore moins d'enquêter systématiquement sur tous ses clients- même lorsqu'aucun indice ne laisse soupçonner l'existence de malversations. Les articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier obligent malheureusement les banques à s'immiscer dans la vie privée de leurs clients. Sous prétexte de lutter contre les « risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme », les banques sont tenues d'obliger leurs clients, au besoin par un chantage à la fermeture du compte, à fournir des détails relevant de leur vie privée, tels que l'état de leur patrimoine et de leurs revenus ou le but de chèques émis, même d'un très petit montant. Cela peut se comprendre pour la souscription d'un emprunt, mais certainement pas pour la simple gestion d'un compte courant, surtout lorsqu'il n'y a aucun indice suspect. Pour parvenir à leurs fins, les banques font croire à leurs clients qu'ils ont l'obligation de répondre, alors qu'aucun texte ne le prévoit. Afin de contourner un Afin de contourner un éventuel refus, le code susvisé permet aux banques de pratiquer un chantage, en menaçant les clients de fermer leur compte. Pire encore, le code permet aux banques de passer outre, même lorsque la Banque de France leur a enjoint d'appliquer le droit au compte. Les conséquences pour les clients en sont exorbitantes, car on ne peut plus vivre normalement dans notre société si l'on n'a pas un compte bancaire. Un tel abus de droit relève du chantage et de l'atteinte à la vie privée. Pire encore, la démarche des banques devient systématique et s'applique même en l'absence du moindre indice laissant soupçonner du blanchiment ou du terrorisme. Afin de garantir le respect de la vie privée de nos citoyens, il faut réagir face à ces pratiques intrusives, qui violent les règles les plus élémentaires de l'État de droit. Il est évident qu'il faut lutter contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme, mais, les banques étant des organismes privés, elles n'ont pas à se charger d'enquêtes policières ou fiscales, notamment lorsqu'il n'y a aucun indice suspect. Si les banques ont des soupçons, la seule procédure respectueuse des libertés publiques est d'alerter les services fiscaux, la justice ou Tracfin.

je ne reviendrai pas longuement sur ce qui a déjà été dit. Il s'agit d'un projet de loi assez technique- technique ne veut pas dire mineur -, qui a été déposé par le Gouvernement pendant la suspension des travaux parlementaires en avril dernier et que la commission des finances a d'ores et déjà examiné selon la procédure de législation en commission, en présence du ministre délégué Jean-Noël Barrot. Autant dire que nous n'avons pas beaucoup eu l'occasion de nous pencher sur ce texte, dont l'examen apparaît comme une quasi-procédure simplifiée. Qu'est-ce que ce livre VII du code monétaire et financier ? Il s'agit du dernier livre de la partie législative de ce code, qui concerne le régime spécifique applicable Les territoires ultramarins se caractérisent par une diversité de statuts juridiques : les cinq départements et régions d'outre-mer, qui sont régis par le principe d'identité législative avec la métropole, à l'inverse de la Nouvelle-Calédonie, qui est une collectivité,

-et disposent de leur propre monnaie, le franc Pacifique, dont le cours, fixé par rapport à l'euro, est d'environ 1 euro pour 120 francs Pacifique- à ne pas confondre avec l'ancienne piastre, qui avait cours à l'époque de l'Indochine Cette diversité de statuts juridiques se traduit dans nos textes par nombre de dispositions spécifiques aux outre-mer. Le présent projet de loi vient d'abord ratifier trois ordonnances, dont celle du 25 février 2022, qui nécessite une ratification impérative avant avant l'été selon la procédure, non pas de l'article 38, mais de l'article 74-1 de la Constitution. J'évoquerai, à cette occasion, le souvenir de l'ordonnance du 9 février 2017 sur l'application du code de commerce en Polynésie française, qui avait déjà fait l'objet d'une loi de ratification adoptée selon cette procédure en 2018. A-t-on eu depuis une évaluation de l'impact de cette ordonnance sur la concurrence et le coût de la vie en Polynésie ? Les dispositions suivantes du projet de loi concernent largement les territoires du Pacifique. À l'article 5, je m'étonne que le retrait d'espèces en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie ne soit gratuit que dans les établissements où l'on détient des comptes, ce qui diffère de la situation en métropole. Y a-t-il une raison précise à cette situation ? Pour le reste, je n'aurai pas de remarque particulière. La situation économique, sociale et politique en outre-mer fait régulièrement l'actualité. Il est aujourd'hui particulièrement question de la situation sécuritaire à Mayotte, avec l'opération Wuambushu, déclenchée le 24 avril dernier.

les récentes élections territoriales en Polynésie ont vu la victoire du camp indépendantiste, tandis que la situation post-référendaire en Nouvelle-Calédonie n'a pas encore débouché sur une solution pérenne. Enfin, dans les Antilles, la situation sociale reste caractérisée par une certaine défiance, alimentée par des scandales comme celui du chlordécone. Le développement socio-économique en outre-mer reste donc une priorité, dans des territoires où le niveau de vie est, en moyenne, le tiers de celui de la métropole. Les territoires ultramarins représentent pourtant une richesse incomparable, à la fois naturelle et culturelle. C'est le premier réservoir de biodiversité en France et un domaine maritime exceptionnel, qu'il convient de préserver face aux effets déjà palpables du changement climatique. le plus possible aux habitants de ces territoires d'être eux-mêmes acteurs de ce développement. En conclusion, mis à part les quelques remarques formulées, le groupe RDSE ne voit pas d'objection particulière à l'adoption de ce projet de loi

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, le présent projet de loi a pour objet de ratifier plusieurs ordonnances relatives à l'outre-mer. Nous nous méfions toujours du recours aux ordonnances, car il dépossède le Parlement de ses prérogatives législatives. Mais, en l'espèce, force est de reconnaître qu'il s'agit de dispositions très techniques, qui ne posent pas de difficultés. Nous resterons cependant extrêmement vigilants. Lors du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, le nombre d'ordonnances avait quasiment doublé. Les ordonnances de septembre 2021, février et septembre 2022, qu'il nous est proposé aujourd'hui de ratifier, ont un double ont un double objet. Tout d'abord, il est proposé d'approuver la recodification du livre VII du code monétaire et financier pour améliorer sa lisibilité. Cette recodification de plus de 500 articles est le fruit d'un long travail, qui a duré trois années. Nous l'approuvons, car l'intelligibilité de la loi était remise en question pour nos compatriotes vivant outre-mer. Il est également proposé de moderniser les missions de l'Institut d'émission d'outre-mer et de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Notre groupe approuve également cette mesure. Nous saluons le travail du rapporteur, Hervé Maurey, qui a permis une amélioration du texte. du texte. La majorité des articles ont été amendés et adoptés la semaine dernière, dans le cadre de la procédure de législation en commission. Parmi les améliorations essentielles, il nous paraît important de souligner que, l'expérimentation visant à ouvrir le financement participatif obligatoire aux collectivités territoriales ayant pris du retard, il était nécessaire de la prolonger de deux ans, afin qu'elle s'effectue sur le temps réellement imparti, soit le délai initial de trois ans. Par ailleurs, concernant la modernisation des missions des Instituts d'émission, la centralisation des informations d'identification des comptes de toute nature sur le même fichier, telle que la propose la commission, nous semble pertinente. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera ce projet de loi, tel qu'il ressort des travaux de notre Haute Assemblée. La parole

étranger. Nous attendons beaucoup de l'opération Wuambushu lancée par le Gouvernement. Paradoxalement, cette situation dramatique apporte aussi des signes d'espoir, puisqu'elle a rappelé à l'ensemble des Français l'attachement sans faille des Mahorais à la communauté nationale. L'État doit se montrer à la hauteur de ces espoirs. L'exemple de Mayotte nous rappelle que, pour consolider l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national, il faut que les lois soient appliquées partout. Toutes proportions gardées, le projet de loi que nous examinons s'inscrit dans cette logique : garantir la bonne application des lois sur l'ensemble du territoire national. Il contient ainsi plusieurs mesures pour adapter le code monétaire et financier aux évolutions récentes. Cela concerne principalement la ratification de trois ordonnances, prises entre septembre 2021 et septembre 2022. Les modifications législatives apportées par ces ordonnances sont essentiellement techniques. Elles n'ont pas déchaîné de débats passionnés au sein de notre commission. Cependant, elles n'en sont pas moins importantes. Elles parachèvent, en effet, un travail de réorganisation législative entrepris il y a plus de quatre ans, au moment de la promulgation de la loi Pacte. Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi réécrit de façon thématique, ce qui rendra notre droit applicable plus lisible. Cette réécriture était, de toute façon, rendue nécessaire par les récentes évolutions législatives, tant au niveau français qu'au niveau Je ne reviens pas sur la méthode retenue pour procéder à la ratification des ordonnances, mais il est vrai qu'il y a toujours quelque chose d'étonnant à présenter une réforme comme urgente alors qu'elle parachève un travail de plusieurs années ... L'essentiel est que nous puissions désormais avancer. Le groupe Les Indépendants - République et Territoires votera en faveur de ce texte. Pour conclure, mes chers collègues, je souhaite évoquer deux amendements adoptés par la commission des finances. Le premier concerne l'article 1. Ce nouvel article prévoit de prolonger l'expérimentation sur l'accès des collectivités au financement participatif. J'ignore si le délai de publication de l'arrêté ministériel révèle quelque réticence de la part de Bercy. Ce que je crois, en revanche, c'est que nous devons donner davantage de libertés aux collectivités, et davantage de moyens aux élus locaux. Il faut faire confiance aux territoires. amendement concerne la suppression de l'article 9, qui visait à donner une base législative au fichier des comptes d'outre-mer (Ficom). J'espère que la navette parlementaire permettra de trouver la solution qui sera à la fois la plus respectueuse des libertés publiques et la plus efficace pour l'ordre public. C'est dans cette tension, mes chers collègues, que nous parviendrons à garantir la cohésion nationale, sur l'ensemble du territoire de la République. La parole

qui est un texte particulièrement technique, un texte de correction rédactionnelle et d'adaptation de fond du code monétaire et financier pour certaines collectivités d'outre-mer, pour lequel je risque de verser dans l'ultracrépidarianisme. Vous connaissez ce terme, qui qualifie un comportement consistant à donner son avis sur des sujets à propos desquels on ne possède pas de compétence crédible ou démontrée. Je remercie d'ailleurs notre collègue Hervé Maurey pour son analyse. Il a rendu ce texte compréhensible et l'a amélioré par ses amendements. Je ne veux pas non plus prendre le risque de dire moins bien que d'autres que l'adoption de ce projet de loi est nécessaire, puisque les ordonnances, dont l'échéance est désormais très proche, doivent être consolidées. Deux mesures contenues dans ce projet de loi appellent notre vigilance.

mérite évidemment d'être retenue. La seconde mesure est la fin de la règle de gratuité totale des retraits d'espèces par carte effectués en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

doit se conjuguer avec la préservation du pouvoir d'achat, moins élevé pour nos concitoyens qui y résident que pour la plupart de ceux qui vivent dans l'Hexagone. À propos des ordonnances, nous ne nions pas leur utilité sur des sujets techniques tels que celui qui nous réunit aujourd'hui. Toutefois, comme le rappelait le président de notre groupe, Guillaume Gontard, lors du débat sur le suivi des ordonnances, en février 2022, « sous le quinquennat Macron, 345 habilitations par ordonnances ont été accordées, et ce nombre a doublé en dix ans- sans doute est-ce d'ailleurs sur ce doublement qu'il faut insister

nous sommes déterminés à ce que ce pouvoir ne soit pas corseté lors des débats qui touchent aux sujets essentiels de la vie de nos concitoyens, comme celui des retraites, et soit peut-être moins sollicité sur des sujets dont la technicité nous éloigne parfois des problèmes les plus essentiels

sérieux. Je pense plutôt à la précarité qui fait rage dans nos territoires, à l'inflation qui frappe plus brutalement les portefeuilles là-bas qu'ici, à la vie chère, au manque d'emplois, à une jeunesse qui manque parfois de perspectives, qui sont le quotidien des habitants des outre-mer. Lorsque je pense aux outre-mer, je pense aussi aux sargasses, à l'orpaillage illégal en Guyane, à la construction controversée de la nouvelle route du littoral à La Réunion, à la défense de la biodiversité des fonds marins, du vivant et des écosystèmes, qui figurent parmi les plus riches au monde et doivent être au coeur de nos actions dans les territoires d'outre-mer, plus encore qu'ailleurs. Je pense également aux batailles juridiques, menées notamment par Harry Durimel, maire écologiste de Pointe-à-Pitre et par d'autres- certains siègent sur nos travées -, pour faire reconnaître les préjudices liés au chlordécone, un scandale sanitaire, social et environnemental

Merci ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer. Mes chers

est suspendue. La séance est reprise. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants

C'est l'objet de la présente proposition de loi, portée avec conviction par M. le député Bruno Studer et, je le rappelle, adoptée à l'unanimité en première lecture par l'Assemblée nationale. L'essor des des réseaux sociaux invite à repenser les moyens de protection pour faire face aux nouvelles dérives qui mettent à mal la vie privée et l'image de nos enfants. Avant l'âge de 13 ans, un enfant apparaît, en moyenne, sur le compte de ses parents ou de ses proches sur 1 300 photographies publiées en ligne. Dans le même temps, les parents d'enfants âgés de moins de 13 ans partagent en moyenne 71 photos et 29 vidéos par an sur les réseaux sociaux. Un cinquième des parents ont des profils Facebook publics, la moitié partagent des photos avec des amis virtuels qu'ils ne connaissent pas vraiment. À cette vitesse, d'ici à la fin de la décennie, les informations partagées en ligne par les parents seront la première cause d'usurpation d'identité pour leurs enfants. Que l'on ne s'y trompe pas : les images des enfants sont bel et bien des données personnelles sensibles, qui soulèvent des enjeux de pédocriminalité, d'identité numérique, d'exploitation commerciale ou encore de harcèlement. Je veux partager avec vous le constat alarmant des auteurs de la présente proposition de loi

Parallèlement, les données personnelles des enfants mises en ligne par leurs parents interrogent les notions de droit à l'oubli et, bien sûr, d'identité numérique. Sur le long terme, mesdames, messieurs les sénateurs, les contenus publiés- même en toute bonne foi -par leurs parents pourraient porter préjudice aux enfants et compromettre, par exemple, leur crédibilité lors d'une candidature scolaire ou professionnelle. Face à ces risques et dans l'intérêt supérieur et bien compris de l'enfant, il est nécessaire de cadrer les conditions d'exercice par les parents de leur autorité parentale en matière de vie privée et de droit à l'image de leurs enfants.

importante dans l'exercice du droit à l'image des enfants exposés sur les réseaux sociaux. Hier même, votre assemblée examinait en première lecture sur une nouvelle proposition de loi visant à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est dire si le monde de l'internet a décidément un grand besoin de régulation, pour les adultes, bien sûr, mais également pour les enfants, en particulier ceux qui n'ont aucune prétention d'être des influenceurs. Cette proposition de loi

L'article 1 modifie l'article 371-1 du code civil afin d'introduire la notion de « vie privée » de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale. À ce sujet, je salue le travail de la commission qui a repositionné l'ajout de la notion de « vie privée » à la fin de l'article 371-1 du code civil : il est plus cohérent de formaliser

Ensuite, il rendait ce droit plus visible pour les parents. Je prends néanmoins acte de la position de la commission sur cet article. L'article 3 a également été modifié pour faire de tous les actes « relatifs à la vie privée de l'enfant » des actes non usuels. Permettez-moi d'exprimer des réserves sur cette nouvelle rédaction. sur son emplacement à l'article 372-2 du code civil. Cet article a, en effet, pour objet de définir le régime juridique de l'acte usuel relatif à la personne de l'enfant et non de de définir ou d'énumérer les actes relevant du régime juridique des actes non usuels. Outre que cette disposition disposition fragilise l'économie générale de l'article 372-2, elle comporte le risque de constituer un précédent en invitant le législateur à dresser une liste des actes usuels et non usuels dans la loi. Or l'établissement d'une telle liste, qui, pour être utile, devrait être exhaustive, n'est en pratique pas possible l'appréciation de ce qui relève d'un acte usuel ou non usuel est nécessairement casuistique. Elle nécessite donc d'être appréciée finement par un juge pour préserver au mieux l'intérêt de l'enfant. Deuxièmement, la notion de « contenus relatifs à la vie privée de l'enfant » est trop large : elle dépasse la publication de la seule image de l'enfant, puisqu'il suffirait que la publication soit relative à la vie privée de l'enfant pour être qualifiée d'acte non usuel et nécessiter alors l'accord des deux parents. Cela induit, à mon sens, un cadre juridique trop contraignant. Surtout, cet article complexifie et rigidifie le quotidien des familles, puisque l'accord des deux parents pourra être systématiquement exigé par les tiers pour toute diffusion de contenu relatif à la vie privée de l'enfant. un tel recueil ne sera pas toujours possible en pratique, par exemple en cas de conflit parental ou d'absence de l'autre parent. C'est cet article instaure surtout une hiérarchie entre les différents droits de l'enfant, au sommet de laquelle se trouverait le droit au respect de sa vie privée. Cela nous semble contestable. Le droit à la vie privée doit-il être plus protégé que le droit à la santé par exemple ? Avec cet article, l'accord des deux parents serait systématiquement exigé pour toute diffusion de « contenus relatifs à la vie privée de l'enfant », alors que, en ce qui concerne la santé de l'enfant par exemple, l'accord d'un seul des parents pourrait, dans certains cas, suffire. Pour toutes ces raisons, je soutiendrai l'amendement de votre collègue Thani Mohamed Soilihi qui permet de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale tout en l'adaptant afin de mieux protéger le droit à l'image des enfants.

utilement la réglementation existante en matière de protection des enfants, notamment en ce qui concerne l'assistance éducative. Votre commission a introduit un nouvel article qui permet à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) de saisir le tribunal judiciaire pour demander en référé le blocage d'un site internet en cas d'atteinte aux droits d'un mineur. Ce dispositif est intéressant, mais devra probablement être réservé aux atteintes les plus graves. Je suis également sensible à l'idée selon laquelle la saisine de la Cnil doit faire suite à la plainte d'un tiers. La navette parlementaire pourra utilement améliorer la rédaction. Face à une exposition accrue des mineurs sur internet et à des risques provenant du foyer familial, il est indispensable de repenser la notion de droit à l'image des enfants et de responsabiliser davantage leurs parents. Je me réjouis donc des débats qui s'annoncent et, vous l'aurez compris, mesdames, messieurs les sénateurs, je soutiendrai cette proposition de loi.

Nous commençons seulement à prendre la mesure des répercussions qu'a sur la santé, le bien-être et le développement de nos enfants un accès potentiellement permanent aux contenus des réseaux sociaux ou des sites internet les smartphones. C'est pourquoi je regrette que ce sujet ne soit pas pris à bras-le-corps par le Gouvernement dans le cadre d'une politique publique nationale réunissant tous les acteurs pouvant agir en la matière. Actuellement, le Sénat est invité à se prononcer sur quatre initiatives visant la protection des mineurs dans l'univers numérique. Outre cette proposition de loi, nous ont été transmises de l'Assemblée nationale, premièrement, une proposition de loi relative à la prévention de l'exposition excessive des enfants aux écrans,

une proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, que le Sénat a adoptée hier soir, dont Mme Amel Gacquerre

... Surtout, une réponse législative n'est pas suffisante : tous les acteurs s'accordent à dire que c'est la prévention, l'éducation et la sensibilisation qui sont efficaces en la matière. S'agissant du sujet qui nous occupe, tous les moyens devraient être mobilisés pour alerter les parents des conséquences d'une diffusion d'images ou, plus généralement, de contenus relatifs à la vie privée de leur enfant dans l'espace numérique en raison des utilisations préjudiciables qui peuvent en être faites par la suite harcèlement scolaire, détournement sur des sites pédocriminels, usurpation d'identité, atteinte à la réputation ... Malheureusement, j'en oublie. Il est particulièrement important que la sensibilisation soit organisée par l'État de manière uniforme sur tout le territoire, car les inégalités en fonction du milieu social sont très importantes en la matière, comme l'ont rappelé la Défenseure des droits et le Défenseur des enfants, que nous avons auditionnés. Pour ma part, je souhaite exprimer trois requêtes au Gouvernement. Ma première demande est la réactualisation du carnet de santé, qui n'a pas été mis à jour depuis 2018

ne peut pas être seulement législative et sectorielle, comme proposé. Elle doit être plus globale. Cependant, la proposition de loi que nous examinons a le mérite de favoriser une prise de conscience collective sur le droit à l'image des enfants. Bruno Studer lui-même l'a décrite comme « une loi de pédagogie à destination des parents. Je pense que nous pouvons souscrire à cet objectif en recentrant cette proposition de loi sur l'essentiel, sans oublier que veiller au respect de la vie privée de l'enfant fait déjà partie de la mission exercée conjointement par les parents dans le cadre de l'autorité parentale, à savoir «

lors des mariages. C'est pourquoi la commission a adopté l'article 1 qui vise à introduire la protection de la vie privée de l'enfant parmi les obligations des parents au titre de l'autorité parentale. Nous en avons préféré la rédaction initiale qui rattache la vie privée de l'enfant au « respect dû à sa personne », sans la placer sur le même plan que la sécurité, la santé et la moralité. En effet, pour assurer ces trois finalités fondamentales, les parents ont un devoir de surveillance dont le degré d'intensité varie selon l'âge, la maturité et la capacité de discernement de l'enfant. Ce devoir peut justifier une atteinte à la vie privée de l'enfant, par exemple pour vérifier avec qui il correspond ou qui il rencontre, dans le but de le protéger. En revanche, la commission a supprimé l'article 2, qui n'est qu'une simple répétition, spécifiquement consacrée au droit à l'image, des dispositions des articles 371-1 et 372 371-1 et 372 du code civil. L'utilisation du code à des fins pédagogiques doit être limitée à l'essentiel. C'est déjà ce que vise l'article 1. À l'article 3, qui n'était qu'un simple rappel du droit existant, nous avons inscrit que « la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l'enfant », ce qui comprend photos et vidéos, nécessite l'« accord de chacun des parents ». Cette disposition éviterait toute divergence d'approche entre juridictions pour décider s'il s'agit d'un acte

Nous avons choisi une formulation large pour inclure toute information relative à la vie privée et couvrir ainsi toute situation, comme la divulgation d'un bulletin de santé. La commission a supprimé l'article 4 qui tendait à permettre une délégation forcée de l'exercice du droit à l'image de l'enfant lorsque la diffusion de l'image de celui-ci porte gravement atteinte à sa dignité ou à son intégrité intégrité morale, ce qu'on appelle les. L'article ne semble en effet pas opérant : en pratique, cette délégation n'aurait que peu d'effet, puisque le parent continuerait à pouvoir filmer ou photographier l'enfant dans son quotidien et poster ces images sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, ce serait mettre sur le même plan des comportements de gravités très différentes, la délégation d'autorité parentale étant réservée au « désintérêt manifeste » des parents, à « l'impossibilité d'exercer tout ou partie de l'autorité parentale » ou au meurtre d'un parent par l'autre. serait un peu curieux. Dans tous les cas, je rappelle que la diffusion d'images de l'enfant « port[ant] gravement atteinte à la dignité ou à l'intégrité morale de celui-ci » caractérise des carences éducatives qui peuvent justifier la saisine du juge des enfants en vue du prononcé de mesures d'assistance éducative. Il n'y a donc pas de vide juridique en la matière, ce qui nous a été confirmé lors de toutes les auditions que nous avons réalisées. Enfin, pour compléter l'article 3 qui pose le principe d'un accord des deux parents pour publier une photo ou une vidéo d'un enfant, la commission a adopté un article 5 permettant à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'agir en référé dès lors qu'il y a une atteinte aux droits des mineurs en matière de données à caractère personnel, sans condition de gravité ou d'immédiateté. La Cnil pourrait sur cette base demander le blocage d'un site internet dont l'éditeur ne répondrait pas aux demandes d'effacement ou ne prouverait pas avoir l'accord des deux parents pour la publication relative à l'enfant.

la numérisation progressive de la société est inéluctable. Qu'on le déplore ou qu'on s'en réjouisse, c'est un fait qui s'impose à nous toutes et à nous tous : nous constatons la multiplication des réseaux sociaux et nous mesurons la massification de leurs usages, pour pour le meilleur et, parfois, pour le pire. Nous sommes toutes et tous susceptibles d'être exposés numériquement, souvent de notre plein gré, mais parfois contre notre volonté. Il en va de même pour les mineurs,

Cela s'est traduit ces dernières années par une multiplication d'initiatives parlementaires visant à faire évoluer notre législation et à l'adapter aux risques d'un genre nouveau. Madame la rapporteure a mis en avant les textes en

Elle permet aux mineurs de demander l'effacement de leurs données personnelles et des images les concernant sans l'accord préalable de leurs parents. Hier, nous étudiions la proposition de loi visant à encadrer l'influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous débattons de la proposition de loi visant à garantir le respect du droit à l'image des enfants. Le 23 mai prochain, nous devrons nous prononcer sur une autre initiative parlementaire, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. Il est à noter que tous ces textes, en tant que propositions de loi, émanent de parlementaires, en l'espèce de députés de la majorité présidentielle. Face aux dangers pouvant être causés par ce nouvel environnement numérique, il est évidemment salutaire que le législateur se saisisse de cette thématique. je rejoindrai là aussi Mme la rapporteure en m'adressant à M. le garde des sceaux : une législation véritablement protectrice ne saurait se bâtir par la multiplication de petites propositions de loi, au champ et à la portée limités, dont les objectifs non coordonnés pourraient être de nature à nuire à la cohérence d'ensemble de notre droit. Ces initiatives parlementaires sont certes les bienvenues, mais force est de constater qu'elles sont partielles et parcellaires. Une fois n'est pas coutume, il nous semble que, pour faire preuve d'efficacité face à un sujet complexe, il eût été préférable que l'exécutif présente un projet de loi transversal et global.

Permettez-moi de rappeler que le dernier texte d'origine gouvernementale date de 2016 et avait été défendu à l'époque par Axelle Lemaire, secrétaire d'État chargée du numérique lors du quinquennat de François Hollande. Ces travaux de Mme Lemaire avaient abouti à l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, comprenant la dernière grande avancée digitale pour les enfants, à savoir une amélioration substantielle du droit à l'oubli des mineurs sur le Net. À l'ère des mutations numériques, 2016, c'est très loin ! c'est très loin ! Depuis, le cyberenvironnement a beaucoup évolué. Les problématiques qui y ont trait se sont encore multipliées, en particulier pour les personnes mineures. Un rapport de 2018 de Mme Rachel de Souza, commissaire à l'enfance pour le Royaume-Uni, peut nous éclairer sur l'ampleur du phénomène dont il est ici question.

Si le fait de poster des photos d'enfants sur les réseaux sociaux peut sembler anodin de prime abord, la situation devient plus grave lorsque celles-ci sont détournées à des fins sordides. Selon les rapports du Centre national pour les enfants disparus ou exploités, qui oeuvre aux États-Unis, la moitié des photographies d'enfants s'échangeant sur les réseaux pédophiles et pédopornographiques ont été à l'origine postées sur le Net par leurs parents, par leur famille ou par leurs proches. Ces publications, innocentes dans l'intention, peuvent donc être source de détournements, mais aussi de cyberharcèlement. Aussi, face à ces risques et à ces dangers aux multiples facettes, nous devons nous interroger sur la pertinence, sur l'utilité et sur l'efficacité du texte que nous étudions aujourd'hui. Il semble que, dans sa forme initiale, cette proposition de loi était dotée d'une portée normative limitée. En effet, ses articles 1, 2 et 3 semblaient relativement superflus, car déjà plus ou moins satisfaits par le droit positif. Tout au plus garantissaient-ils une meilleure lisibilité de notre législation. L'article 4, relatif à la délégation partielle, sous contrainte, de l'autorité parentale, concernait principalement des cas rares, ce qui prédestinait cette mesure à être peu usitée. En raison de ces faiblesses, le texte tel qu'il a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale pouvait davantage être considéré comme une proposition de loi déclarative, visant à sensibiliser l'opinion et notamment les parents aux risques auxquels sont exposés les enfants faisant l'objet de publications sur internet. Déclarer, déclamer, proclamer, c'est bien ; avoir le souci de l'efficacité, c'est mieux. Je sais, madame la rapporteure, que vous avez une appréciation similaire au sujet de cette initiative parlementaire. Vous avez donc souhaité amender ce texte afin d'en garantir une meilleure application et une plus grande efficacité. Je vous en remercie. Cependant, tous les apports et toutes les modifications effectués par la commission ne sont pas de nature à nous convaincre totalement. Nous soutenons évidemment la suppression de l'article 2, dont l'apport n'était pas nécessaire, répétant simplement des dispositions déjà en vigueur dans le droit. Nous nous montrons davantage circonspects quant aux réécritures des articles 1 et 3. Dans les deux cas, il semble que les rédactions choisies puissent donner lieu à interprétation et compliquer, dans la pratique, le travail du juge. Le mérite initial de ces articles était pourtant d'assurer aux professionnels du droit une plus grande clarté de notre législation. Le nouvel article 5 suscite également quelques interrogations. Celui-ci est venu conférer au président de la Cnil, par voie de référé, le droit d'ordonner aux juridictions compétentes toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la vie privée d'un mineur sans que soient requis des critères de gravité ou d'immédiateté, comme c'est le cas actuellement. Le concept même du référé est intrinsèquement lié au caractère urgent d'une situation : il nous semble donc contradictoire d'autoriser une procédure en référé sans que la considération d'urgence du cas d'espèce entre en ligne de compte. De grâce, ne banalisons pas la notion de référé Enfin, nous nous montrons plutôt défavorables à la suppression de l'article 4 de cette proposition de loi. En effet, son dispositif ayant été encadré à l'Assemblée nationale et ne devant concerner que de rares affaires, cette nouvelle mesure aurait pu trouver sa place au sein de notre arsenal législatif. Ces doutes étant exprimés, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain soutiendra malgré tout cette initiative parlementaire. Lacunaire, ne couvrant qu'un pan extrêmement restreint de la thématique que ses auteurs souhaitent traiter, cette proposition de loi ne permettra sans doute pas à elle seule de protéger les mineurs des dangers d'internet. Elle a cependant mérite de mettre en lumière ces nouveaux risques liés à l'univers numérique, en particulier pour les enfants, et elle ouvrira certainement de nouveaux débats en la matière. Aussi, je forme le voeu que le Gouvernement se saisisse pleinement de ce sujet afin que nous puissions rapidement nous doter d'une législation encore plus volontariste et plus protectrice pour toutes et pour tous. La balle est désormais dans le camp de l'exécutif. S'il juge le sujet digne d'intérêt, ce que je crois, il saura saisir l'occasion. La parole est à Mme

collègues, la protection de l'enfant est une question fondamentale- cela a été rappelé -qui doit être constamment prise en compte dans nos sociétés.

avec l'omniprésence des écrans et des réseaux sociaux, l'exposition des enfants sur internet est un phénomène en constante augmentation. Il est de notre responsabilité de moderniser notre législation pour mieux protéger leur vie privée.

seront plus encore à l'avenir si nous n'agissons pas. La rapidité des développements technologiques au cours des dernières décennies a créé de nouveaux défis pour la protection des mineurs. Tout comme l'ont dénoncé la Défenseure des droits et le Défenseur des enfants dans leur dernier rapport annuel sur la protection des droits des enfants, l'utilisation généralisée des écrans et des réseaux sociaux signifie que les enfants sont plus exposés que jamais à des risques tels que le harcèlement en ligne, la cyberintimidation et la violation de leur vie privée. privée. Nous, parents, devons prendre conscience de ces dangers et prendre des mesures pour protéger nos enfants. Nous, législateurs, devons moderniser la loi, y compris le code civil, pour protéger la vie privée des enfants dans le contexte du développement du numérique. Certains pourraient s'inquiéter que des changements dans la loi puissent limiter la liberté des parents d'éduquer leurs enfants comme ils l'entendent. Cependant, il convient de rappeler que l'intention des auteurs de cette proposition de loi n'est pas de restreindre cette liberté, mais plutôt de renforcer la protection des mineurs contre les risques liés à une exposition en ligne. Il est important de souligner que les atteintes à la vie privée des enfants ne sont pas toutes le fait d'intentions malveillantes. Beaucoup n'ont pas conscience des dangers que représentent les réseaux sociaux pour les plus Nous regrettons que la proposition de loi actuelle ne contienne pas de mesures de sensibilisation des parents. Nous devons nous assurer que les intéressés soient pleinement conscients des dangers de publier des photos ou des vidéos de leurs enfants en ligne, même si ces actions sont bien intentionnées. Nous devons les aider à comprendre les risques afin qu'ils prennent des décisions éclairées quant à la façon dont ils exposent leurs enfants.

être résolue par la législation seule. Les entreprises qui fournissent des plateformes en ligne et les réseaux sociaux ont également une responsabilité dans la protection de la vie privée des plus jeunes. Elles doivent mettre en place des politiques efficaces pour prévenir le harcèlement en ligne, la cyberintimidation et la violation de la vie privée de ce public. Elles doivent également s'assurer qu'ils ne soient pas exposés à des contenus inappropriés. Il est crucial que nous ayons une compréhension claire et nuancée de la façon dont les enfants utilisent internet et les réseaux sociaux. Les recherches montrent qu'ils ont souvent des comportements en ligne qui peuvent les exposer à des risques, mais qu'ils sont également capables de gérer ces risques s'ils sont correctement informés. Nous devons également tenir compte des différents âges et du développement des enfants lors de l'élaboration de politiques de protection de la vie privée en ligne, parce que, inévitablement, les problématiques ne sont pas les mêmes.

mes chers collègues, 300 millions, c'est le nombre de photographies qui sont diffusées chaque jour sur les réseaux sociaux. Cette appétence pour le partage de contenus témoigne certainement de la capacité du numérique à créer et entretenir du lien social avec nos proches et nos moins proches. de nos jours, que toute notre activité en ligne, même la plus anodine, est enregistrée, analysée, décortiquée et finalement monétisée. Ces traces, que l'on croyait éphémères et restreintes, sont en réalité visibles par le plus grand nombre et pour longtemps. En outre, on estime qu'un enfant apparaît, en moyenne, sur 1 300 photographies publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, sur ses comptes propres, ceux de ses parents ou de ses proches. Il s'agit de l'un des principaux risques d'atteinte à la vie privée des mineurs, principalement du fait de la difficulté à contrôler la diffusion de son image. En effet, 50 % des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. Pis, les informations diffusées sur le quotidien des enfants peuvent permettre à des individus d'identifier leurs lieux et habitudes de vie à des fins de prédation sexuelle. Enfin, au-delà du risque pédophile, les contenus mis en ligne sont susceptibles de porter préjudice à l'enfant à long terme, sans que celui-ci puisse obtenir leur effacement

d'enjeux économiques forts, à la fois pour les marques, en quête de relais auprès d'un jeune public, et pour les parents. Dès lors, ces derniers doivent assumer un double rôle : celui de gestionnaire et celui de protecteur de l'image de leur enfant. peuvent parfois donner lieu à un arbitrage délicat, car les parents peuvent entrer en conflit avec leur enfant en raison des avantages financiers, sociaux ou émotionnels que l'exploitation de l'image de l'enfant peut apporter. L'enfant peut alors être confronté à un conflit de loyauté entre ses propres aspirations et la volonté de ses parents. D'ailleurs, selon une étude, 40 % des adolescents estiment que leurs parents les exposent trop sur internet. Enfin, l'exposition excessive des enfants au jugement de tiers sur internet et la course aux et autres appréciations peuvent engendrer des problèmes psychologiques, en particulier dans l'acceptation de soi et de son image. Nous voyons parfois les ravages de ce phénomène sur des adultes, alors imaginez sur des enfants le cyberharcèlement y trouve un terreau fécond. Vous l'aurez compris, mes chers collègues, il est utile de légiférer sur ce sujet. Or si le constat dressé apparaît inquiétant et nécessite une intervention de notre part, le texte que nous

En l'état, nous ne pouvons qu'espérer que ce texte suffise. En attendant, notre commission- et je salue le travail de notre rapporteure, Valérie Boyer -a fait le choix d'enrichir et de rendre plus efficace le texte qui nous est proposé, avec pour principal objectif d'éduquer et de sensibiliser les parents. Ainsi, l'article 1 introduit la notion de vie privée de l'enfant dans la définition de l'autorité parentale, pour mieux faire prendre conscience aux parents qu'il leur appartient d'assurer le respect de la vie privée de leur enfant dans le cadre de leur obligation de protection et de préservation de ses intérêts. faisant que reprendre des dispositions déjà consacrées dans le code civil et précisées par l'article 1, notre commission a choisi de le supprimer. L'article 3 précise que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessite l'accord des deux parents,

5 permet à la Cnil de saisir les juridictions compétentes pour demander le blocage d'un site internet en cas d'atteinte aux droits des mineurs. Très bien ! Elle pourra ainsi agir en référé dès lors que les droits de personnes mineures sont concernés, sans condition de gravité ou d'immédiateté de l'atteinte. Tous ceux qui travaillent à protéger les enfants ne peuvent que se réjouir de cette avancée. En conclusion, il s'agit d'un texte pédagogique et de prévention que le groupe Union Centriste votera.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la moitié des photographies échangées sur les réseaux pédopornographiques avaient initialement été publiées sur les réseaux sociaux ce n'est pas le seul danger auquel sont exposés ces enfants : mises en scène dégradantes pour faire rire, influenceurs qui font commerce de leur vie de famille ... Ces pratiques favorisent le Ces pratiques favorisent le harcèlement scolaire et les problèmes liés à l'intimité, l'acceptation de soi et de son image. Un enfant apparaît en moyenne sur 1 300 photos publiées avant l'âge de 13 ans, alors qu'il n'a pas encore la maturité nécessaire

Ce texte ouvre la voie à des relations conflictuelles aussi bien entre les parents et leurs enfants qu'entre les parents eux-mêmes. eux-mêmes. Le respect de la vie privée de l'enfant devant toujours rester notre priorité, des propositions complémentaires seraient nécessaires afin de mieux sensibiliser aux conséquences de cet exercice du droit à l'image. Lorsque cette image est exploitée par des parents qui en font leur fonds de commerce, peut-être serait-il juste, par exemple, que ces enfants perçoivent une rémunération appropriée à leur majorité. Si nous ne devons pas nous satisfaire de cette proposition de loi, elle a toutefois le mérite de poser les fondements d'une protection du droit à l'image des enfants. La parole

charrie des risques n'épargnant pas les plus jeunes. Nous pensons, par exemple, au cyberharcèlement ou à la collecte de données. Il va sans dire que la protection de l'enfance intéresse, naturellement, le Sénat- et la commission des lois en particulier -au-delà de la seule question des nouvelles technologies.

Comme nous l'avions souligné dès les premières lignes de ce rapport d'information : « Les violences sur mineurs, qu'elles soient de nature physique, sexuelle ou psychologique, ou les privations qui leur sont infligées, parce qu'elles concernent les plus fragiles d'entre nous, sont devenues insupportables dans notre société.

Ce n'est évidemment pas le cas, car, d'une part, rien n'est léger quand il est question des plus jeunes et, d'autre part, l'ampleur des difficultés rencontrées avec le numérique ne doit pas être sous-estimée.

de questions particulièrement complexes touchant, au fond, toutes les générations. D'ailleurs, la Cnil nous alerte depuis plusieurs années sur ces sujets et nous incite à prendre en compte le point de vue et les droits de l'enfant dans la conception des services et l'élaboration des réglementations. faut aussi protéger les enfants contre l'exploitation commerciale de leurs données. De même, nous devons soutenir le rôle fondamental d'accompagnement des parents et des acteurs de l'éducation.

introduire la notion de vie privée dans la définition de l'autorité parentale soulignera l'importance que les parents doivent accorder à cette question, au même titre qu'ils doivent veiller à la sécurité, à la santé ou à la moralité de leur enfant. D'aucuns doutent qu'une telle disposition puisse produire des effets efficaces et concrets, mais elle indique la bonne démarche. De la même manière, la nouvelle rédaction de l'article 3 semble satisfaisante : la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée de l'enfant devra être l'objet d'un accord de chacun des parents.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la protection des mineurs dans un univers numérique devenu omniprésent constitue un défi majeur pour notre société. Il s'agit d'un enjeu à la fois pour les familles, en premier lieu les parents, et pour les institutions, en matière d'éducation et de santé publique. À l'heure où les réseaux sociaux inondent notre quotidien, plus de 300 millions de photos y étant diffusées chaque jour, et où le est devenu une valeur de référence, le phénomène de surexposition sur internet est une réalité. Cette réalité présente de multiples dangers, souvent pas

rappelle que la moitié des images qui se trouvent sur les sites pédopornographiques avaient été initialement publiées par les parents. Par ailleurs, en moyenne, avant l'âge de 13 ans un enfant apparaît sur 1 300 photographies publiées en ligne, et un tiers des enfants ont une existence sur internet avant même d'être nés.

prise en considération. Au reste, l'examen de la jurisprudence nous démontre que cette question est déjà soumise aux juridictions, notamment en cas de conflit entre les parents. Je salue le travail mené par la commission des lois, en particulier par notre collègue rapporteure Valérie Boyer, dont je sais l'engagement de longue date sur le sujet. Comme l'a indiqué cette dernière, la vocation de ce texte est avant tout pédagogique, afin de sensibiliser, informer et alerter les parents sur les dangers que peut présenter un tel affichage de leur enfant. Les parents appartenant de plus en plus à une génération du tout-numérique, le partage des photos peut leur paraître anodin

pédagogique que pour son réel apport juridique. Mais voyons en ce texte une première étape, car sans pédagogie, sans explication et sans information, aucune politique publique ne peut être efficace. C'est d'autant plus vrai que les parents sont les premiers éducateurs des enfants.

de mener une véritable politique publique en la matière. En ce sens, je partage l'avis de notre rapporteure, dont le travail a également permis de formuler des recommandations que je salue, notamment la création d'une page dans le carnet de santé sur l'exposition aux écrans. Par une approche constructive du texte, la commission a choisi d'intégrer

que son respect incombe déjà aux parents dans le cadre de l'autorité parentale. De même, j'approuve la suppression par la commission de l'article 2, puisque le droit à l'image est d'ores et déjà exercé en commun

de l'article 3 de manière à inscrire dans la loi que la diffusion de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessite l'accord des deux parents évitera des interprétations multiples sur la

puisse solliciter le blocage d'un site internet qui ne répondrait pas aux demandes d'effacement. Très bien ! Mettre en lumière le respect de la vie privée des mineurs, c'est aussi sensibiliser les jeunes eux-mêmes. Je rappelle que 63 % des moins de 13 ans ont un compte sur un réseau social et que 80 % des parents déclarent ne pas savoir exactement ce que leurs enfants y font. Sensibiliser les parents revient donc à sensibiliser également les enfants, qui sont de futurs ou d'actuels utilisateurs des réseaux sociaux. En conclusion, ce texte met en évidence un problème émergent, mais pourtant déjà bien ancré dans notre société, qui nécessite de trouver un point d'équilibre entre, d'une part, la liberté d'expression des parents

-Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le développement de l'usage du numérique présente bien des avantages, notamment en permettant de conserver un lien social et familial malgré la distance géographique. La diffusion de photographies de famille ou de vidéos sur les réseaux sociaux remplace nos anciens albums photos. Une fête de famille, des vacances, des loisirs, un événement sportif ou culturel, la fête de l'école ... : tout est prétexte à partager la vie de ses enfants. Or si la généralisation de l'usage d'internet et des réseaux sociaux dans nos vies a fait émerger de nouvelles opportunités, elle expose également nos concitoyens à de nouveaux risques et menaces que nous devons prendre en En effet, dans le cyberespace, ces photos, ces vidéos, ces renseignements personnels peuvent être visualisés et repartagés à l'insu des intéressés. Ainsi, la moitié des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques auraient été initialement publiées par les parents sur les réseaux sociaux. sociaux. Ces derniers diffusent bien souvent des photos et des vidéos de leurs enfants sans penser à tous ces risques ; il est urgent de mieux les informer ! Aussi, en raison de la surexposition grandissante de l'image de l'enfant et de l'usage malveillant qui pourrait en être fait par des tiers, il semble primordial d'adapter notre arsenal juridique pour mieux appréhender l'exercice des droits des enfants dans cet environnement numérique. La proposition de loi que nous examinons cet après-midi ne réglera pas tous les problèmes. Elle ne rendra pas non plus à certains parents le bon sens qui leur manque, mais elle permettra sensibilisation et responsabilisation des parents pour protéger les droits des enfants. En faisant oeuvre de pédagogie, elle aura le mérite de rappeler à tous que l'enfant n'est pas un objet, mais une personne titulaire de droits fondamentaux pour sa propre construction, comme le droit à l'image. Lors de l'examen du texte en commission, des modifications utiles et pertinentes ont été apportées. Je rejoins la position de la commission, qui a consacré de façon expresse l'obligation des parents de veiller au respect de la vie privée de leur enfant, y compris de son droit à l'image, au titre de leurs prérogatives liées à l'exercice de l'autorité parentale. Je me réjouis également que la commission ait souhaité que la diffusion au public d'images relatives à la vie privée d'un enfant- photos ou vidéos -nécessite l'accord des deux parents. je me félicite que la commission ait renforcé le pouvoir de la Cnil en cas d'atteinte aux droits des mineurs. Ainsi, celle-ci pourra agir en demandant de bloquer un site internet dans les cas où l'éditeur ne répondrait pas aux demandes d'effacement ou ne prouverait pas avoir obtenu l'accord des deux parents pour la publication concernant l'enfant. Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, à l'ère de l'ultra-digitalisation, les enfants sont plus que jamais mis en danger par leur surexposition sur internet, particulièrement sur les réseaux sociaux. Il est donc nécessaire que nous nous accordions sur un texte opérant, afin de continuer à garantir à l'ensemble des mineurs une protection suffisante. Le groupe Les Indépendants accompagnera toute démarche tendant à préserver les intérêts de l'enfant. Avec conviction, il votera en faveur de cette proposition de loi, utilement modifiée en commission. La parole

constante et à coût constant a démocratisé l'accès au numérique, au point que nous avons désormais toutes et tous des téléphones portables, des iPads- comme celui sur lequel je lis mon intervention -, des ordinateurs, qui nous permettent de tout photographier, de filmer chaque moment de la vie et de les partager en direct sur les réseaux sociaux.

est-il évident qu'il nous faut mieux encadrer le droit à l'image des enfants dans la loi pour enfin tenir compte de la démocratisation du numérique et de l'exposition des mineurs. C'est pourquoi le groupe écologiste soutient

Cette disposition vient utilement compléter une proposition de loi qui comportait jusque-là un angle mort : au-delà des mesures visant à responsabiliser les parents, la responsabilité des opérateurs de réseaux sociaux avait été quelque peu oubliée. Pourtant, les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans les atteintes au droit à l'image des enfants. ces images sont-elles diffusées ? Elles ne sont pas placardées dans la rue ; elles sont publiées sur les réseaux sociaux ! En complément du droit à l'oubli, qui permet aux enfants ou aux enfants devenus majeurs de demander le retrait de ces publications- il s'agit d'un élément très important nous souhaitons permettre aux titulaires de l'autorité parentale de demander le retrait d'images montrant leurs enfants diffusées par des tiers. Concrètement, le groupe écologiste demande que tout opérateur d'un réseau social mette en place un mécanisme de signalement afin que les parents puissent signaler des images de leurs enfants ayant été diffusées sans ou contre

Un enfant peut être gêné par une photo et exprimer une opposition à sa publication en ligne ; il faut en tenir compte. Ce n'est pas facile à faire : j'ai moi-même fait l'expérience de tenter d'expliquer ce qu'implique la publication d'une photo sur les réseaux sociaux à ma nièce de 6 ans. Il s'agissait d'un dessin qu'elle avait fait.

avant de publier une image, et même lorsqu'ils le font, tous n'ont pas conscience de l'importance de cette demande ni de la manière de la formuler. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons inscrire dans la loi le fait que les parents doivent associer leurs enfants à l'exercice du droit à leur image en fonction de leur âge et de leur degré de maturité. Au fond, la réponse au développement du numérique

l'essor du numérique et l'avènement des réseaux sociaux ont profondément révolutionné la vision que nous avons de notre image et l'usage que nous en faisons pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. Dans ce contexte, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui tend à mieux faire respecter le droit à l'image des enfants par leurs parents, qui en sont responsables. Cela a été répété, mais il faut le redire, à l'âge de 13 ans, un enfant a déjà en moyenne 1 300 images de lui qui circulent sur internet Ce comportement numérique des parents, apparemment anodin, n'est pourtant pas dénué de risques. Ces risques sont d'abord pédocriminels, puisque 50 % des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées par les parents sur leurs réseaux sociaux. ensuite liés à la prédation sexuelle, car les lieux fréquentés par les enfants ou les informations personnelles qu'ils livrent peuvent être identifiés sur des photos. Des risques de cyberharcèlement, de harcèlement scolaire ou encore d'usurpation d'identité, enfin, peuvent aussi exister. Évidemment, l'immense majorité des parents agit par naïveté. La fierté et la méconnaissance des dangers liés au partage de l'image de leur enfant sur internet les poussent parfois à l'imprudence. Quelques-uns le font par bêtise, malveillance ou profit. C'est pourquoi il était nécessaire d'essayer de trouver un équilibre entre liberté d'expression et intérêt supérieur de l'enfant, entre sensibilisation aux risques et répression. Ce texte, à visée pédagogique surtout, s'inscrit dans la droite ligne de plusieurs initiatives parlementaires qui ont été prises au cours des dernières années en vue de renforcer la protection du droit à l'image des enfants sur internet. Je pense notamment à la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui a reconnu aux mineurs un droit à l'oubli numérique, à la loi du 19 octobre 2020 visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne, grâce à laquelle les mineurs n'ont pas besoin du consentement de leurs parents pour demander l'effacement de leurs données personnelles.

également engagé à accompagner les parents face aux enjeux de parentalité numérique pour prévenir les usages excessifs et inappropriés des écrans, en soutenant ces initiatives parlementaires, en lançant une campagne nationale de prévention consacrée à la parentalité numérique ou encore au travers de la création d'une plateforme d'information et d'accompagnement à la parentalité numérique. Plus précisément, la proposition de loi qui est soumise

en revanche, choisi de supprimer l'article 2, qu'elle a jugé redondant, et l'article 4, dont les dispositions ont été considérées comme inopérantes.

toute image de son enfant sans l'autorisation de l'autre parent lorsqu'il y avait désaccord entre eux sur l'exercice des actes non usuels relevant du droit à l'image de l'enfant. Afin d'éviter une interprétation différente de la notion d'actes usuels ou non usuels entre juridictions, la commission a décidé d'inscrire dans la loi que la diffusion au public de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant nécessiterait l'accord des deux parents et et que, en cas d'atteinte aux droits des mineurs en matière de données à caractère personnel, la Cnil pourrait agir en référé. Il nous semble important de renforcer la protection des enfants tout en évitant de rigidifier à l'excès le quotidien des familles, ce que, à notre sens, cette nouvelle rédaction risque de provoquer. Aussi, nous vous soumettrons un amendement proposant de permettre au juge d'interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent, sans faire référence aux actes non usuels de l'autorité parentale qui figurait dans le texte adopté par l'Assemblée nationale. Le groupe RDPI se félicite de l'examen de ce texte qui répond à un défi sociétal actuel et accompagnera les parents dans l'exercice de leur parentalité numérique, afin d'éviter un usage abusif du droit à l'image des enfants et leur surexposition sur les plateformes sociales.

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le développement des réseaux sociaux et leur utilisation massive par un public jeune et moins jeune ont créé une situation d'immersion massive de nos enfants dans l'espace numérique. Nous n'avons pas fini de découvrir ce nouveau continent, qui a ses espoirs, mais aussi ses travers. Ce n'est pas la première fois que le législateur ou les pouvoirs publics interviennent dans le champ numérique par rapport aux enfants. Dans le passé, nous avons réagi au au phénomène de cyberharcèlement ; récemment, nous l'avons fait sur les enfants influenceurs et sur la majorité numérique. On le voit, nous sommes véritablement au coeur d'une préoccupation qui touche tous les éducateurs, tous les parents. Internet peut en effet donner le meilleur comme le pire. Le romantisme des ou l'innocence des ne doivent pas occulter ce sombre terrain de chasse pour les prédateurs et autres usagers malveillants. Les chiffres sont terrifiants. Plus de 300 millions de photographies sont diffusées par jour sur les réseaux sociaux, 1 300 photographies par enfant sont publiées en ligne avant l'âge de 13 ans, 50 % des photographies qui s'échangent sur les forums pédopornographiques ont été initialement publiées par les parents sur les réseaux sociaux- sans oublier les nombreuses images détournées. Dans ce souci de protéger les plus fragiles, nous devons donc préserver le droit à l'image des enfants, des enfants exposés, trop exposés. Le respect du droit à l'image n'est au fond qu'une application des exigences de l'autorité parentale qui s'imposent aux parents au titre de l'article 371-1 du code civil, que beaucoup de ceux qui, parmi nous, ont été officiers d'état civil comme maires ou adjoints au maire connaissent.

C'est aussi la pratique par certains parents du, ces canulars aux dépens de l'enfant, qui peuvent provoquer chez ce dernier des troubles psychologiques altérant l'acceptation de soi et de son image. En effet, c'est d'abord aux parents qu'incombe la protection de leurs enfants dans cet univers numérique. La solution est donc dans ces obligations qui s'imposent aux parents au nom de l'exercice de l'autorité parentale. Puisqu'ils veillent à la sécurité et à la santé de leurs enfants dans le respect dû à leur personne, comme l'affirme le code civil, les parents doivent en tirer toutes les conséquences. Aux parents de limiter l'exposition des enfants aux écrans. Cela a été dit, mais cela doit être encore rappelé. Il faut fixer des limites et éviter une familiarisation précoce aux écrans. C'est un enjeu de santé et de sécurité dans la protection des enfants. Rien ne pourra remplacer la responsabilité des parents, qui est immense dans ce domaine Aux parents eux-mêmes de faire preuve de sobriété en évitant de communiquer des photos ou des vidéos où l'on voit leurs enfants. Cette sobriété numérique doit profiter à tout le monde et respecter l'intimité de l'enfant, surtout à un moment où les vies privées sont encore liées et, dans tous les sens du terme, connectées. C'est par ailleurs pour cette raison que la commission des lois a préféré une rédaction plus modeste de l'article 1 du texte pour tenir compte du fait que la sécurité, la santé et la moralité peuvent justifier une atteinte à la vie privée de l'enfant Cette obligation de veiller au respect de la vie privée de l'enfant s'inscrit dans l'exercice de l'autorité parentale. Parce que l'enfant est encore sous la dépendance de ses parents, même s'il publie souvent seul les photos, la commission des lois a rappelé le nécessaire accord des deux parents pour la diffusion au public de contenus relatifs la vie privée de l'enfant. Cela permet de rappeler la gravité de cet acte, donc de mieux réfléchir à la publication de ces images. Cela permettra aussi d'éviter des divergences éventuelles entre juridictions, par exemple sur l'autorisation de l'un ou des deux parents pour publier une image. des parents divorcés pas toujours en accord ? Si la protection du droit à l'image des enfants revient aux deux parents, encore faut-il les aider dans cette tâche lourde et pourtant noble. Au-delà de l'utilité ou de la pertinence de tel dispositif dans notre législation, nous souffrons surtout de l'absence d'une véritable politique publique de l'espace numérique. Toutes les familles ne sont pas logées à la même enseigne et la prévention reste encore un domaine lacunaire. Il faut une véritable politique globale, et non une simple réaction au coup par coup. Certes, rien ne remplace les parents, mais on peut tout de même les aider et les accompagner. Il faut une aide à la parentalité dans ce domaine, comme nous le voyons au travers de certaines initiatives de terrain. La société, l'école ont aussi un rôle à jouer. L'information à l'égard des parents doit être développée. Ils sont les premiers garants de la protection de leurs enfants et doivent être alertés notamment sur la conséquence de la diffusion d'images. La santé doit aussi englober le volet numérique. Il faut en effet parler de « santé numérique », laquelle reste évidemment dans le prolongement de la santé physique ou mentale, mais tend tout de même à devenir un domaine spécifique. Il faut utiliser les vecteurs traditionnels et les adapter à ce nouveau contexte. Dans son rapport, notre collègue Valérie Boyer préconise la création d'une nouvelle page dans le carnet de santé, qui pourrait contenir des informations sur l'exposition des enfants aux écrans ou aux réseaux sociaux. Parce qu'il n'y a pas de prévention sans mise en cause des dangers, il faut élaborer un véritable programme de santé publique, qui doit accompagner tous les enfants dans leur parcours scolaire, et ce de la maternelle au lycée. Dans toutes les étapes de leur scolarité, les enfants doivent, dès leur plus jeune âge, être sensibilisés aux risques d'internet, afin que leur droit à l'image soit préservé. Plus ce sera tôt, mieux ce sera, et ce de la manière la plus pédagogique possible. Ce que nous avons fait contre la drogue ou contre l'obésité, nous pouvons le faire sur l'usage d'internet et sur celui des réseaux sociaux. N'ayons pas peur de sensibiliser les enfants et de leur parler des dangers auxquels ils sont exposés. C'est toujours en le disant que les choses vont mieux ! N'attendons pas des drames et ne nous résignons pas à rester les bras croisés au prétexte que l'on ne peut pas faire grand-chose dans cet univers complexe. La fluidité d'internet ne saurait justifier l'absence d'interdits ni surtout d'appréhension des conséquences pérennes de ces diverses publications, tout comme l'absence du droit à l'oubli. Le passé numérique ne doit pas devenir Monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, le défi est vaste, mais les enfants sont l'avenir de notre société et nous devons à tout prix les préserver ! L'impératif de protection doit l'emporter quand il s'agit de la jeunesse. Le groupe Les Républicains votera en faveur de cette proposition de loi.

En commission, l'article 3 a été entièrement réécrit : désormais, la diffusion publique de contenus relatifs à la vie privée d'un enfant est subordonnée à l'accord des deux parents. Si nous saluons la volonté de la rapporteure de créer les conditions d'une harmonisation de la jurisprudence, nous craignons que la notion très large de « contenus relatifs à la vie privée de l'enfant » ne complexifie le quotidien des familles. En effet, la rédaction retenue par la commission aurait notamment pour conséquence d'obliger les tiers à recueillir l'accord des deux parents pour les diffusions restreintes et conformes à l'intérêt de l'enfant, par exemple dans le cadre scolaire. Par ailleurs, nous considérons que le dispositif proposé par la commission tend à instaurer une hiérarchie injustifiée entre les différents droits de l'enfant. Il entraînerait en effet une sanctuarisation du droit à la vie privée, alors que, pour les actes concernant d'autres droits, tels que le droit à la santé, l'accord d'un seul parent pourrait suffire. toutes ces raisons, nous proposons de rétablir le texte adopté par l'Assemblée nationale, tout en supprimant la référence aux actes non usuels de l'autorité parentale. Concrètement, nous proposons d'accorder au juge la possibilité d'interdire à un parent de diffuser tout contenu relatif à son enfant, sans l'autorisation de l'autre parent en cas de désaccord sur l'exercice du droit à l'image de l'enfant. Cette interdiction concernerait à la fois les actes usuels et les actes non usuels de l'autorité parentale.

de saisir le juge aux affaires familiales, y compris en référé, pour solliciter l'interdiction de diffuser tout contenu relatif à l'enfant. J'y suis favorable, parce que, dans un contexte d'exposition accrue accrue de l'image des enfants, ce que nous déplorons tous, il me semble tout à fait important de rappeler que le juge aux affaires familiales peut interdire la diffusion d'images d'enfants.

explication de vote. J'ai entendu les explications de Mme la rapporteure : il est vrai que le sujet mérite d'être encore travaillé.

la publication reste visible jusqu'à l'aboutissement éventuel d'une procédure de demande de retrait et elle peut être partagée. Cela a été dit, de nombreuses photos se retrouvent ainsi sur des sites pédocriminels et on ne peut pas faire comme si ce n'était pas un danger majeur. D'autre part, cela exclut des enfants plus jeunes qui pourraient dire non à leurs parents, mais qui seraient, de fait, incapables de remplir un formulaire pour demander le retrait d'une photo déjà publiée. de donner plus de droits aux enfants, nous proposons de rétablir une disposition qui a été supprimée en commission. Plus concrètement, il s'agit de demander aux parents d'associer l'enfant à l'exercice de son droit à l'image. J'ai bien conscience que l'on ne peut pas facilement associer un enfant de 2 ans à l'exercice de son droit à l'image. Pour autant, c'est possible pour une adolescente de 14 ans. C'est la raison pour laquelle

satisfait déjà les précautions que vous que vous souhaitez prendre, madame la sénatrice Vogel.

ici, quel que soit le mérite de ces structures, c'est à l'État de prendre en charge cette question sur la base d'un programme qui soit identique sur tout le territoire. Si l'on parle bien de démocratie numérique,

quelques instants. La séance est suspendue. En application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution, ainsi que de la loi organique et de la loi ordinaire du 23 juillet 2010 prises pour son application, la commission des affaires sociales a émis, lors de sa réunion de ce jour, un avis favorable- 20 voix pour, 2 voix contre -à la nomination de M. Jean-François Delfraissy à la présidence du Comité consultatif national d'éthique. Par ailleurs, en application des mêmes dispositions, la commission de l'aménagement du territoire a émis un avis défavorable- 8 voix pour, 28 voix contre -à la nomination de M. Marc Papinutti à la présidence de la Commission nationale du débat public. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire

Bien que le célèbre papier rose à trois volets ait laissé place à un nouveau format, commun à tous les pays de l'Union européenne, son caractère primordial reste inchangé. Nous partageons tous- j'en suis convaincue -le constat qu'il s'agit d'un sujet essentiel, au coeur des préoccupations de tous les Français. Toutefois, le Gouvernement n'ignore pas que la préparation à cet examen se révèle parfois laborieuse et est encore bien trop souvent freinée par des enjeux de coûts et de délais. Afin de lever de tels obstacles, le permis de conduire a fait l'objet de réformes ambitieuses, engagées par le Président de la République. La loi du 6 août 2015 a permis de réduire de manière significative les délais d'obtention du permis de conduire grâce à l'externalisation de son épreuve théorique. Dans cette même dynamique, le Gouvernement a présenté en 2019 un plan « pour un permis pour tous, moins cher et plus rapide », avec dix mesures pour réformer le permis de conduire. figuraient des modes d'apprentissage plus modernes, moins chers et plus rapides, comme le simulateur de conduite, l'apprentissage avec une boîte automatique, mais aussi l'encouragement à la conduite accompagnée ou supervisée. En 2021, la plateforme RdvPermis a révolutionné le processus d'attribution des places à l'examen en responsabilisant davantage les candidats. À l'heure de dresser le bilan, force est de constater que les délais d'attente, bien que diminués, demeurent aujourd'hui encore un obstacle dans l'obtention du permis de conduire. La présente proposition de loi, portée par la majorité présidentielle et adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 mars dernier, a pour objectif de poursuivre le travail de modernisation. Elle est le fruit d'un travail de terrain, au plus près des préoccupations de nos concitoyens et des difficultés que peuvent rencontrer, notamment, les jeunes. L'article 1 vise à créer une nouvelle plateforme numérique, « 1 jeune, 1 permis », recensant l'intégralité des aides mises en oeuvre par l'État et les collectivités territoriales pour financer le passage du permis de conduire. Le coût moyen du permis en France est de 1 592 euros. Pour alléger la charge que peut représenter son financement, différentes aides publiques existent, mais leur visibilité reste limitée par la dispersion de l'information. La plateforme « 1 jeune, 1 permis » y remédiera. Pôle Pôle emploi a déjà développé une plateforme, mes-aides.pole-emploi.fr, orientée vers les demandeurs d'emploi et recensant les aides et conditions d'éligibilité des collectivités territoriales ayant transmis volontairement ces informations. Afin de limiter les coûts d'investissements et de capitaliser sur la visibilité de la plateforme, le Gouvernement proposera un amendement visant à en confier la gestion à Pôle emploi, qui deviendra prochainement France Travail. Travail. Il engagera des travaux pour l'améliorer et la rendre accessible depuis un nouveau portail, « 1 jeune, 1 permis », afin de ne pas limiter l'information au public des seuls demandeurs d'emploi et de gagner en visibilité auprès de tous les publics, et notamment des jeunes. L'article 1 prévoit que la préparation et le passage de l'épreuve théorique pourront être organisés hors temps scolaire dans les locaux des établissements scolaires. Cet apport du député Pierre Henriet facilitera les conditions de préparation à l'examen pour nos jeunes. nos jeunes. Face au frein que représente le coût du passage de l'examen du permis de conduire, l'article 2 prévoit d'étendre les possibilités d'utilisation du compte personnel de formation (CPF) à toutes les catégories de permis. La prise

Le Gouvernement espère que cet élargissement constituera un outil précieux d'autonomie et d'insertion professionnelle. Un des ultimes freins à l'obtention du permis est aussi le manque d'examinateurs et le nombre insuffisant de places pour l'examen pratique qui en découle. du ministère de l'intérieur (Lopmi), vous avez acté le recrutement exceptionnel de 100 inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière supplémentaires sur quatre ans. Cela permettra déjà d'accroître durablement l'offre d'examens.

Notre boussole demeure l'accès au permis de conduire pour tous. Nous nous sommes engagés auprès de la députée Piron à trouver des solutions concrètes face aux difficultés de certains jeunes ayant quitté le système scolaire français pour obtenir l'attestation de sécurité routière (ASR). Les solutions identifiées, auxquelles nous associerons les parlementaires, passeront par la voie réglementaire. Enfin, nous connaissons tous les préjugés, parfois sexistes, qui pèsent lorsque l'on parle de permis de conduire. Je connais l'engagement des deux rapporteurs sur les enjeux d'égalité femmes-hommes. Le Gouvernement continuera d'apporter son entier soutien aux travaux qui pourraient être menés sur le sujet. Lever les obstacles au passage du permis de conduire, c'est favoriser la mobilité de nos jeunes, contribuer au désenclavement des territoires les plus éloignés et soutenir l'accès des actifs à un outil essentiel. Lever les obstacles au passage du permis de conduire, c'est garantir l'émancipation, aussi bien personnelle que professionnelle, des Français. Lever les obstacles au passage du permis de conduire, c'est agir concrètement sur le quotidien des Français. La parole

du permis de conduire. Vous l'avez souligné, madame la secrétaire d'État, le permis de conduire est le premier examen de France. Il attire plus d'un million et demi de candidats chaque année et demeure un élément structurant de notre société. Il permet de se déplacer, mais aussi, bien souvent, d'accéder à un emploi. Cependant, le dispositif coûte très cher. D'abord, le coût moyen du passage du permis de conduire est de 1 592 euros, ce qui correspond à une durée moyenne de formation de près de trente heures pour un prix horaire moyen de 53 euros. une fois l'examen obtenu, l'achat et l'entretien du véhicule représentent également des sommes importantes. C'est la raison pour laquelle une réflexion a été engagée depuis quelques années sur les moyens de réduire le coût du passage du permis de conduire. La loi du du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités ont tenté de réduire les coûts d'obtention et de diminuer les délais de passage des examens pratiques et théoriques. Plus ces délais sont longs, plus les candidats sont amenés à prendre des heures supplémentaires de conduite pour maintenir leur niveau, et, au final, plus le coût est élevé. La proposition de loi de notre collègue Sacha Houlié s'inscrit dans cette perspective et a pour objectif de faire face à deux difficultés majeures dans le passage du permis de conduire : le coût et les délais d'obtention. Il s'agit en premier lieu de faire mieux connaître et de renforcer les aides disponibles pour l'apprentissage de la conduite. En ce sens, l'article 1 vise à recenser sur une plateforme unique l'ensemble des aides financières existantes à la préparation des examens du code de la route et du permis de conduire. Cette plateforme permettrait de s'assurer de la contribution de l'ensemble des financeurs du permis de conduire, renforçant ainsi l'accessibilité des aides proposées.

Cela me semble être une bonne idée ; cette proposition paraît plus pratique que le texte initial. Afin de renforcer les aides disponibles pour la formation à la conduite, l'article 2 de la proposition de loi prévoit de rendre éligible au CPF la préparation du code de la route de l'épreuve pratique de l'ensemble des catégories de permis de conduire à compter du 1 janvier prochain. Seraient ajoutés à la situation actuelle les permis motos, voiturettes et remorques. La commission des lois y a souscrit, et je vous propose de faire de même en séance. Il faut cependant souligner que les concertations qui seront conduites avec les partenaires sociaux devront répondre à deux enjeux forts : la soutenabilité financière de cette extension et la préservation d'un lien avec l'emploi dans les dispositifs financés par le CPF. Le troisième enjeu Le troisième enjeu du financement du permis de conduire par le CPF est celui de la lutte contre la fraude. C'est justement à celui-ci que propose de répondre l'article 2 , qui rendrait destinataire la Caisse des dépôts, dépôts, gestionnaire du CPF, des informations relatives au permis de conduire. Cet ajout lui permettra de vérifier que les personnes souscrivant à un financement du CPF sont bien celles qui passent l'examen.

est d'améliorer les délais de passage des épreuves du permis de conduire. L'article 3 étend à l'ensemble des départements le recours aux agents publics ou contractuels comme examinateurs des épreuves de conduite. Ce recours n'est aujourd'hui possible que dans les départements où le délai médian entre deux présentations à l'épreuve pratique du permis de conduire est supérieur à quarante-cinq jours. Cet élargissement permettra d'affecter des examinateurs dans des départements où le délai médian, même s'il est modéré, cache une situation de tension sur les effectifs des inspecteurs. La rédaction proposée transformait cependant une obligation en une simple possibilité à la main du Gouvernement. La commission des lois a donc complété la rédaction de l'article, afin qu'un effort particulier de recrutement soit réalisé dans les départements où le délai de présentation au permis de conduire est excessif. Il est vrai que nous ne

L'Assemblée nationale a également souhaité simplifier la procédure permettant d'organiser dans les lycées, en dehors du temps scolaire, l'épreuve théorique du permis de conduire, et l'élargir à la préparation de cette même épreuve. C'est l'article 1 de la proposition de loi. La simplification proposée conduisait à écarter complètement la collectivité propriétaire, à savoir le conseil régional, de la décision d'occupation des locaux. Nous avons décidé de la réintégrer.

Je vous proposerai également, par un amendement portant article additionnel, d'aligner les peines encourues en cas d'agression sur un examinateur du code de la route sur celles encourues en cas d'agression sur un inspecteur du permis de conduire. Il convient en effet de mieux protéger les examinateurs pour s'assurer du bon fonctionnement de ces épreuves, qui sont désormais souvent externalisées. Enfin, l'Assemblée nationale a adopté deux demandes de rapport. La première concernait le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre du passage de l'examen du permis de conduire. Nous avons obtenu des chiffres, et nous les avons fait figurer dans le rapport de la commission. Il existe un écart notable dans les taux de réussite aux examens théorique et pratique du permis de conduire entre les femmes et les hommes.

La seconde demande concerne l'abaissement de l'âge d'obtention du permis de conduire. Cela s'inscrit dans le cadre de réflexions actuellement conduites par le Gouvernement, qui envisage la création d'un permis provisoire limité au cadre professionnel, sur le modèle d'un dispositif existant en

pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Que fait un étudiant face à cela ? Un chômeur qui doit absolument obtenir le permis ? Le smicard qui compte ses fins de mois, encore plus dans une situation de crise ? Et j'en passe

ou répondre aux besoins personnels. Le droit à la mobilité est un réel sujet, auquel il faut apporter des solutions concrètes pour que les Français et les Françaises puissent s'émanciper, être autonomes et construire sereinement leur parcours de vie.

d'aggraver les inégalités sociales et territoriales dans notre pays. Nous aurions pu, là encore, nous attendre, dans le cadre d'une semaine réservée par priorité au Gouvernement, à un véritable projet de loi, visant à répondre à ces défis.

En effet, il existe de nombreux dispositifs d'aide pour le financement du permis de conduire. Ce texte permettra de rendre plus lisibles les aides des collectivités territoriales en créant une plateforme numérique. Pourquoi pas ?

Nous le verrons dans les années à venir. L'emploi d'agents publics contractuels permettra-t-il réellement de réduire les délais de passage ? Nous le verrons dans les années à venir. Comme nous ne nous opposons pas à cette volonté de relever les défis, nous voterons cette proposition de loi.

Si, pour les urbains, les transports en commun sont un bon moyen de déplacement, pour les ruraux, la voiture individuelle reste souvent la seule option disponible. Ainsi, pour les jeunes, l'obtention du permis de conduire est le sésame vers l'émancipation et l'autonomie. C'est un prérequis indispensable à l'insertion professionnelle. Le permis de conduire constitue le premier examen de France, avec plus d'un million et demi de candidats chaque année. Pourtant, l'âge moyen d'obtention augmente ; il est aujourd'hui de 23 ans. La principale raison d'un tel désintérêt réside probablement dans le coût d'obtention. Certes, le permis de conduire n'a jamais été peu coûteux, mais il faut aujourd'hui débourser entre 1 600 euros et 2 000 euros pour l'obtenir, et ce avec de fortes disparités territoriales. Les délais à rallonge pour passer l'examen sont aussi une cause de surcoût, les candidats étant naturellement amenés à prendre plus d'heures de conduite, sans que cela garantisse la réussite à l'examen. Le taux de réussite, qui est en baisse par rapport aux années précédentes, n'est que de 58,7 % à l'examen de conduite, et de 50,2 % au code. 50,2 % au code. Exact ! Dans l'Yonne, il y a malheureusement un certain nombre de jeunes qui, après avoir été décrocheurs scolaires, sont en grande difficulté pour trouver du travail. L'une de ces difficultés réside dans l'absence de permis de conduire et de véhicule. La plupart du temps, ils ont essayé de passer le permis, et ont échoué au code

au mieux un scooter, au pire une voiture. Et lorsqu'ils se font arrêter sans permis, on leur demande de se rendre au tribunal, à 50 kilomètres de là, sans transport en commun ... Une telle situation n'est pas satisfaisante

nos auto-écoles ... Mais ce texte n'est pas totalement dépourvu d'intérêt ; il contient même des mesures de bon sens. Dans le détail, l'article 1 prévoit la création d'une plateforme recensant l'intégralité des aides disponibles pour la préparation du permis de conduire. Oui, il existe des aides pour financer son permis de conduire. La délégation à la sécurité routière ne recense pas moins de douze dispositifs départementaux et plus d'une centaine de dispositifs communaux ou intercommunaux. Beaucoup d'aides donc, sans doute un peu trop pour que l'aspirant conducteur s'y retrouve. La création de cette plateforme nationale sera donc un précieux outil, de nature réglementaire bien sûr, mais utile. Notre commission- je salue ici le travail et l'enthousiasme de notre rapporteur, Loïc Hervé -a fait le choix de supprimer une disposition adoptée en séance à l'Assemblée nationale : il était prévu que les collectivités et structures apportant un financement aux candidats pour le permis de conduire établissent chaque année un bilan de leurs interventions. probablement la meilleure façon de les dégoûter d'aider ! Sinon, dans ce texte, l'article 1 vise à simplifier le cadre juridique permettant d'organiser dans les lycées, en dehors du temps scolaire, l'épreuve théorique du permis de conduire et sa préparation, en se contentant de l'autorisation du représentant de l'établissement.

Enfin, l'article 3 étend les possibilités de recourir aux agents publics comme examinateurs des épreuves de conduite du permis B, en supprimant la condition limitant cette possibilité aux seuls départements où le délai médian entre deux présentations d'un même candidat est supérieur à

le 14 août prochain, nous fêterons les 130 ans du décret du préfet Lépine aux termes duquel nul « ne pourra conduire un véhicule à moteur mécanique s'il n'est porteur d'un certificat » pour lequel il aura fait « la preuve, devant l'ingénieur en chef des mines chargé du service des appareils à vapeur, qu'il possède l'expérience nécessaire pour l'emploi prompt et sûr des appareils de mise en marche et d'arrêt et pour la direction du véhicule ». Cette première à Paris allait se généraliser moins de dix ans plus tard. Ce bref détour historique nous rappelle combien le sujet du permis de conduire n'a rien d'anodin. La question de son obtention est primordiale, notamment dans les territoires ruraux, où la voiture reste pour les habitants le meilleur, si ce n'est le seul, moyen de déplacement. La problématique peut se décliner de plusieurs manières. Une première est celle des carences en matière de mobilité collective. Dans de nombreux territoires, les transports en commun sont encore trop peu développés. À l'heure où chacun scrute son bilan carbone, à l'heure où le prix de l'énergie et des carburants s'envole, l'État doit donner les moyens aux Français de vivre, en recourant le moins possible à la voiture individuelle. La tâche a été réalisée dans les grandes villes et souvent de manière réussie. Le chantier est d'envergure dans le milieu rural et souvent impossible. Malgré tout, il faut continuer d'avancer. du permis de conduire nous pousse aussi à réfléchir aux problématiques de sécurité routière. C'est d'ailleurs l'essence de ce certificat de capacité qu'avait institué le préfet Lépine. Après une tendance à la baisse au début des années 2010, nous observons une stagnation des chiffres de l'accidentalité routière dans notre pays. Sans surprise, les touchés, notamment par les accidents mortels, sont les jeunes conducteurs, en particulier ceux âgés de 18 ans à 25 ans. Il y a évidemment une part d'inéluctable dans ce constat : l'inexpérience des novices. Mais il existe certainement des axes d'amélioration. Cela peut venir des outils pédagogiques comme du développement de la conduite accompagnée, mais également des campagnes de sensibilisation ou du renforcement des sanctions, notamment en ce qui concerne l'alcoolémie ou la consommation de stupéfiants. Enfin, s'interroger sur l'obtention du permis de conduire revient à s'interroger sur son coût et sur l'accès à l'examen. Nous arrivons ici au coeur de cette proposition de loi, qui ne sera peut-être pas la plus révolutionnaire et la plus attendue de la législature, mais qui aborde une difficulté que rencontre chaque jeune majeur. Si l'on en croit une étude récente, le coût moyen du permis de conduire en France est de 1 804 euros lorsqu'il est passé dans une auto-école traditionnelle. C'est un montant évidemment important, surtout lorsqu'on le demande à quelqu'un qui doit aussi financer ses études, voire un logement. Tout le monde n'a pas la chance de pouvoir compter sur ses parents pour tout cela. Bien entendu, comme l'ont souligné les auteurs du texte, il existe de nombreux dispositifs d'aide pour le financement, comme le permis à un euro par jour pour les jeunes, l'aide financière pour certaines personnes inscrites à Pôle emploi ou encore la mobilisation du compte personnel de formation pour certains permis. Je ne vois donc aucune difficulté à la mise en place d'une plateforme numérique nationale d'information sur les dispositifs de financement du permis de conduire, même si je ne suis pas sûre qu'une loi soit nécessaire pour cela. Je rejoins la position de notre commission, qui, sur l'initiative de son rapporteur, a supprimé l'obligation de bilan annuel, trop lourde et peu utile, pour les collectivités et structures apportant un financement.

cela ne me semble pas être une solution pérenne. Il existe un corps de métier spécifique, celui des inspecteurs du permis de conduire, qui suivent un parcours et une formation adaptés. Nous pensons qu'il vaudrait mieux valoriser ce métier et recruter davantage d'inspecteurs plutôt que de participer à une tendance à laquelle notre groupe n'est pas favorable : l'augmentation du nombre des agents contractuels dans la fonction publique.

il était hier un sésame incontournable et convoité ; il est désormais boudé pour son coût, sa difficulté et une utilité jugée moindre. Le permis de conduire, qui a fêté son centenaire l'année passée, se heurte aux aléas de notre époque. D'abord, les contraintes liées à la sécurité routière ont amplement complexifié son obtention, notamment en zone urbaine. On dénotait ainsi 47 % de réussite à l'examen pratique dans le Rhône ou à Paris contre 75 % en Lozère ou encore 78 % à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ensuite, son coût a considérablement augmenté : de 1 500 francs en moyenne, soit 200 euros, en 1981 contre 1 592 euros en moyenne en 2022, là encore, avec de grandes disparités territoriales. Enfin, le développement des nouvelles mobilités ou les considérations écologiques rendent son obtention moins nécessaire qu'elle ne l'était par le passé, notamment pour les résidents des zones urbaines. Pourtant, le permis de conduire demeure le passeport vers la liberté pour un grand nombre de jeunes au lendemain de leurs 18 ans. C'est le seul moyen pour nombre de nos concitoyens d'assurer leur autonomie dans les territoires ruraux ou les petites villes, où l'offre de transports est souvent insuffisante, voire inexistante. Il est par ailleurs indispensable au quotidien à la mobilité de millions de travailleurs, au point d'être une condition de recrutement sur certains emplois. C'est pourquoi il paraît aujourd'hui quasiment anachronique que le permis de conduire demeure un parcours du combattant pour autant de personnes : 20 % des Français en âge de travailler, soit 7 millions d'individus, se trouveraient en situation de précarité en 28 % des personnes en insertion professionnelle auraient même déclaré avoir dû refuser une formation ou un emploi en l'absence de moyens de déplacement. Il convient bien évidemment de saluer l'initiative de cette proposition de loi. Les rectifications apportées par notre collègue rapporteur, Loïc Hervé, vont dans le sens d'un assouplissement des contraintes techniques et administratives qui pèsent sur l'examen. Je pense plus spécifiquement à la suppression du bilan mentionné à l'article 1, qui imposait aux collectivités de retracer l'ensemble des financements apportés aux candidats au permis. L'objectif de transparence est louable ; imposer une nouvelle contrainte sur les collectivités ou les missions locales l'est moins. Je salue aussi la suppression de l'article introduit par les députés qui tendait à renvoyer à un décret en Conseil d'État la tâche d'assouplir l'exigence de présenter l'ASR ou l'ASSR 2 pour les moins de 21 ans. Cependant, il reste plusieurs points sur lesquels le texte ne répond pas pleinement aux problématiques identifiées sur le sujet. Le recrutement de nouveaux inspecteurs du permis par voie externe est une première avancée, mais elle ne saurait résoudre durablement la question des délais de présentation de l'examen, quand on sait que les facteurs susceptibles de prolonger ceux-ci sont davantage d'ordre financier pour bon nombre de nos concitoyens. Le financement par le CPF est une solution judicieuse pour les personnes en emploi. La proposition d'une cessibilité au sein d'un seul et même foyer, comme entre parents et enfants, est le fruit d'une bonne intention, mais devra être retravaillée pour combler les risques de fraude et de mésusage et pour atténuer les risques d'iniquité. Les droits à la formation sont en effet variables selon la profession, généralement plus généreux pour les professions les plus qualifiées. Cela risquerait donc de pénaliser les ménages les moins aisés. Le principal problème réside, sans surprise, dans le coût de l'épreuve et des heures de conduite. Les aides financières sont insuffisantes et cette proposition de loi n'y apporte pas de solutions concrètes. Les missions locales pour l'emploi et la formation, les centres communaux d'action sociale (CCAS) et les agences de Pôle emploi peuvent apporter un complément de financement pour aider les plus en difficulté, mais elles ont des moyens d'action limités. Le plan gouvernemental « 1 jeune, 1 solution » devra aller plus loin sur les financements proposés et associer les collectivités dans le pilotage de ces fonds. Enfin, je ne suis pas favorable à un abaissement trop important de l'âge légal d'obtention du permis. On a pu observer dans les dernières statistiques fournies par que la mortalité décroissait avec l'âge : le ratio moyen atteint 101 tués par million d'habitants pour les jeunes de 18-24 ans, avant de descendre à 61 pour les 25-34 ans, puis à 52 pour les 35-74 ans. Si un abaissement de l'âge venait à être adopté, il faudrait absolument mettre les bouchées doubles sur la sensibilisation et la prévention routières dans les collèges et les lycées. À l'heure actuelle, les campagnes font effet, mais elles ne sont pas encore suffisantes.

pour faire du permis de conduire une étape accessible à tous financièrement et matériellement, tout en gardant comme finalité suprême la lutte pour la sécurité routière. Le groupe Les Républicains votera cette proposition de loi, mais appelle le Gouvernement à consolider les moyens de son action en la matière. La parole

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, chaque année, 1,5 million de nos concitoyens aspirent à obtenir leur permis de conduire, un rite de passage vers l'indépendance et la mobilité. Cependant, les candidats se heurtent à des obstacles financiers et à des difficultés pour obtenir des heures de formation ou un créneau pour l'examen pratique. Si le permis demeure pour les plus jeunes une première étape vers davantage d'autonomie, c'est aussi un passeport incontournable pour l'emploi, ainsi qu'un outil primordial de l'insertion sociale, en particulier dans les territoires ruraux. Je le mesure dans les 207 communes de mon département. Cette réalité justifie que le législateur cherche à lever les obstacles qui freinent l'accès au permis de conduire, afin de permettre à tous les candidats de se présenter à l'examen dans des conditions de délai et de coût raisonnables. La proposition de loi que nous examinons ce soir tend ainsi à faciliter le passage et l'obtention de l'examen du permis de conduire. Ce texte s'articule autour de trois objectifs : rendre l'accès au permis moins coûteux, plus simple et plus rapide. L'article 1 a pour objet la création d'une plateforme numérique unifiée destinée à rassembler toutes les aides financières accessibles aux jeunes pour les accompagner dans l'obtention de leur permis de conduire. Cette initiative revêt une importance cruciale, car elle vise à offrir une visibilité nationale et simplifiée sur les soutiens disponibles de la part tant des collectivités territoriales que de l'État. Trop souvent, nos jeunes concitoyens se voient contraints d'abandonner leur projet de préparation au permis en raison du coût moyen de 1 600 euros qui peut représenter un obstacle insurmontable pour certains. En facilitant l'accès aux aides existantes, cette plateforme numérique incarne un véritable enjeu d'égalité des chances permettant à chaque jeune de bénéficier d'un accompagnement adapté pour franchir cette étape déterminante de sa vie. L'article 1 vise, quant à lui, à simplifier la procédure permettant d'organiser la préparation et le passage de l'épreuve théorique dans les établissements scolaires. Il présente présente une indéniable utilité, car il renforce l'accès au permis de conduire, notamment pour les élèves des zones rurales souvent délaissés et éloignés des écoles de conduite et des centres d'examen. d'examen. L'article 2, en étendant le financement du permis de conduire à toutes les catégories grâce au compte personnel de formation, offre une nouvelle perspective aux personnes en quête d'emploi. Plus de la moitié de celles qui ont utilisé leur CPF pour obtenir leur permis ont vu leur situation professionnelle s'améliorer. Le permis de conduire est un véritable levier pour redonner confiance pour redonner confiance et espoir à ceux qui cherchent un emploi, en leur permettant de surmonter les obstacles et d'accéder à de nouvelles perspectives professionnelles. L'article 2 procède à l'ajout de la Caisse des dépôts et consignations, de sa mission de gestion du système d'information du CPF, à la liste des autorités, organismes et agents auxquels sont communiquées les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis afin de protéger l'intégrité du permis et de combattre les fraudes. L'enjeu de l'article 3 est de réduire le délai entre deux passages de l'examen. L'élargissement des postes d'examinateur à d'autres catégories d'agents publics pallie le manque d'inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, mais peut susciter une inquiétude catégorielle. Enfin, l'article 3 apparaît intéressant, en prévoyant la remise d'un rapport du Gouvernement au Parlement qui permettra d'analyser les conséquences d'un éventuel abaissement de l'âge d'obtention du permis de conduire.

Cela peut être à l'origine de nouvelles fraudes qui peuvent avoir pour conséquence des retraits de points et de permis pour des personnes victimes de plaques dupliquées.

mes chers collègues, dans les territoires ruraux, les petites villes et les montagnes, la mobilité passe inévitablement par le permis de conduire, qui constitue un passeport pour l'embauche, les visites du quotidien, les loisirs ou encore la vie sociale. et Territoires partage évidemment la volonté de faciliter le passage et l'obtention du permis de conduire et votera, vous l'aurez compris, en faveur de cette proposition de loi.

est d'abord une question de justice sociale. L'un des freins à l'obtention du permis de conduire est son coût, et il n'est pas juste que cela soit facile pour certains et beaucoup plus difficile pour d'autres. En particulier quand on est jeune, la

Monsieur le président, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, au nom du groupe RDPI, je tiens tout d'abord à saluer l'excellent travail de notre rapporteur, Loïc Hervé. Nous souscrivons pleinement aux modifications qu'il a proposé d'apporter au texte adopté par l'Assemblée nationale et porté par les députés Aurore Bergé et Sacha Houlié. Le permis de conduire est souvent qualifié de précieux sésame. Cette expression n'est pas galvaudée, bien au contraire. En effet, pour de nombreux jeunes, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales et périurbaines, le permis de conduire constitue, plus que jamais, un passeport vers l'autonomie personnelle et professionnelle. Chacun de nous se souvient probablement de l'émotion ressentie au moment de la remise du fameux « papier rose » à l'issue de l'épreuve pratique.

Elle a eu pour effet d'allonger les délais d'attente. Ainsi, en 2021, le délai d'attente médian pour un candidat entre sa première et sa deuxième présentation à l'examen pratique du permis B était de

Le texte soumis à notre examen est donc bienvenu. Plus de 100 ans après la création du permis de conduire, il apparaît nécessaire de faciliter le passage de ce permis, qui est le premier examen de France en volume.

Vous l'avez indiqué, madame la secrétaire d'État, c'est une liberté essentielle à la mobilité sociale et professionnelle. Selon nous, le texte dont nous sommes saisis participe de la concrétisation de la promesse républicaine d'émancipation portée par le Président de la République depuis 2017. de renforcer l'accessibilité de l'information relative au financement du permis de conduire, d'élargir les possibilités de financement par le compte personnel de formation et de faciliter le recours à des agents publics ou contractuels en tant qu'examinateurs, en plus du recrutement de 100 inspecteurs supplémentaires d'ici à 2025. Toutes ces dispositions vont dans le bon sens. Elles viennent utilement compléter la réforme déployée par le Gouvernement depuis 2019. Le périmètre du texte est relativement restreint- vous en conviendrez, monsieur le rapporteur -, et je souhaite élargir quelque peu notre discussion. peu notre discussion. Le permis de conduire est synonyme d'émancipation pour nos concitoyens les plus jeunes, d'autonomie bien sûr, mais aussi de responsabilité, et ce à tout âge de la vie. Je tiens à insister sur ce point, car j'ai récemment eu l'occasion de recueillir le témoignage poignant d'une jeune sportive, Pauline Déroulède. Voilà quelques années, elle a été fauchée par un conducteur très âgé qui a perdu le contrôle de sa voiture et a accéléré au lieu de freiner. Malheureusement, elle a perdu sa jambe sur le coup, et sa vie a radicalement changé.

Je vous parlais, mes chers collègues, d'autonomie et de responsabilité. Il ne s'agit pas ici de discriminer les personnes les plus âgées ni même d'envisager de leur retirer un vecteur d'autonomie. Mais, trop régulièrement, des drames de ce genre font la une des journaux et nous ramènent au même débat, sans apporter de réponses concrètes. C'est pourquoi j'invite tous les parlementaires qui souhaitent se pencher sur la question à explorer de nouvelles pistes en vue de prévenir la survenance de ce genre d'accident de la route. L'instauration de visites médicales obligatoires, qui auraient lieu régulièrement tout au long de la vie, est une piste possible. Ces examens permettraient de valider l'aptitude des conducteurs. De nombreux

de loi, qui doit nous réunir, sans clivage, car elle concerne un grand nombre de nos concitoyens. Réduire le coût et les délais de passage du permis de conduire, c'est finalement améliorer la mobilité, favoriser le désenclavement des territoires ruraux et faciliter l'accès des actifs à un outil souvent indispensable. Pour conclure, j'aimerais rappeler que, si la mobilité pour tous est un droit, nous devons accorder une attention accrue aux publics les plus précaires,

La première consiste en la création d'une plateforme numérique nationale recensant l'intégralité des aides distribuées par l'État, les collectivités territoriales et leurs groupements à destination des particuliers. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ne peut qu'approuver l'objectif d'une meilleure information de nos concitoyens potentiellement éligibles à ces aides. C'est de nature à diminuer les inégalités et à augmenter le recours à ces aides. En commission, nous avons d'ailleurs contribué à améliorer le dispositif qui nous était proposé, en insistant sur la nécessité de mettre à jour ces informations. Nous avons de même renvoyé explicitement au pouvoir réglementaire le soin de préciser quels services de l'État seront responsables de la gestion et du suivi de la nouvelle plateforme numérique.

Nous savons à quel point le coût du permis de conduire représente une dépense importante pour un grand nombre de Françaises et de Français, alors même que la détention d'un permis de conduire de catégorie B est bien souvent une nécessité pour entrer sur le marché du travail. Ce permis de conduire est un levier utile pour l'insertion tant professionnelle que sociale. Aussi, nous saluons l'amendement de nos collègues écologistes tendant à la remise d'un rapport gouvernemental sur les possibilités de création d'un service public gratuit de l'enseignement théorique du permis de conduire de catégorie B. Nous comprenons le sens de cet amendement d'appel,

l'article 1 , on crée la possibilité de préparer et de passer l'épreuve théorique du permis de conduire dans les locaux des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté. Le rapporteur Loïc Hervé, que je veux saluer à cette occasion, a amélioré la rédaction du dispositif, tout en maintenant son contrôle par la collectivité propriétaire des locaux. Nous aurions toutefois aussi souhaité recueillir l'avis du conseil d'administration de l'établissement, l'auteur de cette mesure de simplification adoptée à l'Assemblée nationale ayant avancé qu'elle s'inscrivait dans un objectif pédagogique global porté par l'établissement. Le conseiller régional d'Occitanie que je suis ne peut que souscrire à une telle analyse et, par conséquent, regretter que la disposition n'ait pas été retenue. Le périmètre de certaines aides au passage de l'examen de conduite du permis de conduire est actuellement trop restreint, en particulier s'agissant du compte personnel de formation, alors même que l'on connaît l'importance que revêt l'obtention du permis, quelle que soit sa catégorie, dans la recherche d'un travail. Nous ne pouvons donc qu'approuver le dispositif prévu à l'article 2, qui étend les possibilités d'utilisation du CPF à toutes les catégories du permis de conduire, ainsi qu'à la préparation théorique de ces épreuves.

Aussi, l'article 3 légèrement modifié par le rapporteur, permettrait l'externalisation de certaines missions de manière à compléter les effectifs des inspecteurs. Si nous partageons le constat, nous ne soutenons pas nécessairement la solution apportée. Comme ma collègue Maryse Carrère, je considère qu'il y a toujours mieux à faire que de recourir à des contractuels pour

L'automobile, rappelons-le, n'est ni un luxe ni un plaisir futile : c'est d'abord un outil indispensable dans la vie quotidienne de nos concitoyens. L'apprentissage de la conduite est une démarche complexe, qui reste très souvent à la charge de celui ou de celle qui envisage de conduire. Les coûts en sont élevés, même si beaucoup a été fait pour faciliter l'accès au permis de conduire et que les collectivités locales, souvent pionnières dans ce domaine, sont impliquées. Néanmoins, en général, pour obtenir le fameux sésame, il faut débourser- les chiffres ont déjà été cités -autour de 1 500 euros. Les prix des leçons

par quelques solutions pratiques. Cela passe d'abord par l'information. L'absence de visibilité des dispositifs de financement laisse trop de nos concitoyens dans l'ignorance. Aussi sera mise en place une plateforme numérique, destinée à faire connaître les dispositifs de financement de la formation à la conduite que l'État, les collectivités locales ou toute autre structure publique seront susceptibles de proposer aux particuliers. Cette plateforme devra également permettre de choisir son établissement de conduite et de s'inscrire à l'examen du permis. Je m'étonne que cela n'ait pas été fait plus tôt, alors que le numérique occupe une place croissante dans nos vies. Honneur au Parlement d'avoir pris les devants et proposé un dispositif officiel d'information à la charge de l'administration ! Se pose ensuite la question de la formation. C'est aussi un volet complexe, car l'apprentissage de la conduite demande des sacrifices financiers, mais aussi de son temps et de ses déplacements. Il faut faciliter la vie de ceux qui veulent passer le code de la route. Cela passe par un meilleur appui aux jeunes, qui se destinent forcément à une vie professionnelle. Aussi, ce texte permet que la préparation et le passage de l'épreuve théorique soient organisés dans les locaux des lycées et des établissements régionaux d'enseignement adapté. C'est reconnaître que les établissements d'enseignement sont appelés à être des lieux de formation.

Il faudra donc davantage aider ce jeune public désireux d'acquérir un instrument précieux pour son autonomie, mais aussi réfléchir à une meilleure formation au permis de conduire sur tous les lieux de travail ou d'apprentissage à la vie professionnelle.

voire sur son avenir même, on avait peut-être oublié qu'il existait des formations indispensables à privilégier. L'apprentissage de la conduite en est une. Mieux vaut tard que jamais ! Cela donnera également plus de visibilité au CPF, qui n'est pas toujours connu et qui semble encore compliqué à utiliser. Enfin, ce texte est le fruit de travaux effectués par les parlementaires. Il a été précédé par plusieurs études et observations faites sur le terrain, dans le cadre tant de la fonction législative que de la mission de contrôle de nos assemblées. Cette proposition de loi démontre que le législateur peut, après un minutieux travail d'évaluation, se saisir des sujets du quotidien et proposer des solutions pratiques, un exemple qui doit être poursuivi dans d'autres domaines.

J'ai cependant été très étonné, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, que trop peu de cas soit fait des taux de réussite à l'examen, ainsi que des moyens de les augmenter, dans les réflexions qui nous conduisent à examiner ce texte aujourd'hui. Ce taux n'est que de 57 % à l'échelle nationale, et même de 52 % seulement dans mon département ; c'est bien cette double réalité qui m'a conduit à m'intéresser au sujet et à chercher des solutions. À ce titre, la conduite accompagnée présente bien des avantages. D'abord, elle permet de mieux former et préparer à l'examen de conduite, puisque 3 000 kilomètres doivent être parcourus.

premier lieu, de dresser un bilan du dispositif en vigueur depuis l'arrêté du 16 juillet 2019, qui « a ouvert la possibilité de se présenter à l'examen pratique du permis de conduire dès l'âge de 17 ans pour les candidats ayant choisi une formation en conduite accompagnée, afin de pouvoir commencer à conduire en autonomie dès le premier jour du 18 du 18 anniversaire », comme il est très bien rappelé dans le rapport de la commission. Alors qu'en Meurthe-et-Moselle, seuls 25 % des jeunes ont recours à la conduite accompagnée, ce qui est déjà un très bon score, ce rapport aurait permis de mieux comprendre les motivations et les freins à l'engagement dans cette procédure. cette procédure. Je suggérais également que le Gouvernement, à l'occasion de ce rapport, se penche sur l'opportunité de créer un vivier d'accompagnateurs bénévoles pour accompagner les jeunes dont le foyer n'a pas de voiture, ou dont les parents n'ont pas le permis ou la disponibilité nécessaire pour effectuer les 3 000 kilomètres kilomètres dans le temps imparti. Même si, dans les faits, l'accompagnateur à la conduite accompagnée peut être choisi hors du cadre familial du jeune, la quasi-totalité des accompagnateurs sont les parents ou, éventuellement, les grands-parents, ce qui est logique.

permis B depuis plus de cinq ans, accord de l'assurance automobile, absence d'annulation ou d'invalidation du permis dans les cinq années précédentes, etc. La création de ce vivier officiel de bénévoles, qui pourrait même être labélisé, serait une partie de la solution aux problèmes et aux freins que rencontrent ces jeunes et leurs familles.

mon amendement, je profite de cette intervention pour vous proposer de mener à bien cette démarche, ou du moins d'expérimenter cette création d'un vivier dans quelques départements, en lien avec les missions locales et avec l'ensemble des acteurs qui interviennent sur les questions de jeunesse. Ce n'est pas dans cet hémicycle, mes chers collègues, que je vais vous apprendre à quel point le permis de conduire est un sésame indispensable à la vie quotidienne ! La discussion

est à Mme la secrétaire d'État. L'article 1 de cette proposition de loi vise à mieux faire connaître les aides actuellement disponibles pour financer le permis de conduire. Elles sont nombreuses et ont différentes origines- régions, départements, communes -, mais elles ne sont pas toujours lisibles. C'est pour y remédier qu'est prévue, à cet article, la mise en place d'une plateforme unique recensant l'ensemble de ces aides financières. Or il existe déjà une plateforme qui remplit ce rôle

et les services de Pôle emploi. Le présent amendement vise à capitaliser sur cette plateforme existante et sur la visibilité qu'elle a déjà acquise, en confiant la gestion de la future plateforme de recensement des aides à cet opérateur majeur du ministère du travail. Bien entendu, comme l'objectif est de s'adresser à tous les publics et non pas uniquement aux demandeurs d'emploi, Pôle emploi fera évoluer la plateforme actuelle.

Il convient de relever que confier la gestion de cette plateforme à Pôle emploi fait particulièrement sens dans le cadre de la mise en place de France Travail. Ainsi, grâce à la gouvernance partagée entre l'État et les collectivités territoriales, le recueil d'information et l'actualisation des aides mises en place dans les territoires seront facilités. C'est une chose de disposer d'une plateforme ; la maintenir

et de la sécurité routière (IPCSR) dans leur mission principale, celle d'examinateurs de l'examen pratique du permis B, ce qui permettra de réduire les délais d'attente pour le passage de l'épreuve pratique du permis de conduire. L'article 3 ne vise en aucun cas à remplacer les inspecteurs du permis de conduire ou à faire disparaître leur corps. Au contraire, ce dispositif favorise même le recrutement d'agents supplémentaires : ainsi, trente-huit des agents de La Poste recrutés en tant qu'examinateurs ont choisi leur intégration dans le corps des IPCSR.

M. le rapporteur. Cet amendement vise à faire bénéficier les examinateurs des centres organisant, pour le compte de l'État, le passage de l'examen du code de la route ou des épreuves pratiques des permis de conduire de véhicules du groupe lourd de la même protection

du Gouvernement ? Effectivement, les examinateurs de l'épreuve théorique générale et les examinateurs agents publics ou contractuels chargés des examens pratiques de la catégorie B, qui ont pour mission d'assurer le respect des règles de passage de ces épreuves,

et de la sécurité routière. La modification ici proposée à ces articles permettra de sanctionner les agresseurs de ces examinateurs de l'interdiction administrative de se présenter à l'examen du permis de conduire pour une durée de deux à six mois, en anticipation de la peine complémentaire judiciaire d'interdiction de se présenter à l'examen pour une durée de trois ans ou plus. Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Comment répondre à l'injustice entre ceux qui peuvent bénéficier de la conduite accompagnée et ceux qui ne le peuvent pas, parce que leur foyer n'a pas de voiture ou que leurs parents n'ont pas le permis ou la disponibilité nécessaire pour effectuer les 3 000 kilomètres requis dans le temps imparti ? Que pensez-vous de ma proposition de création d'un vivier d'accompagnateurs bénévoles, par exemple des pompiers ou gendarmes retraités, qui pourraient être labélisés, pour aider les jeunes ? C'est une idée que je défends depuis quelques mois, grâce au remarquable travail d'un stagiaire de troisième accueilli l'année dernière, Sacha Vettese, qui est présent dans nos Après nos rendez-vous avec le préfet de Meurthe-et-Moselle et la générale de gendarmerie déléguée à la sécurité routière, Florence Guillaume, il nous apparaît qu'une telle idée est vraiment à creuser et qu'il y a matière à expérimenter. Elle apporterait une partie de la solution aux problèmes et aux freins que rencontrent les jeunes et leurs familles. Je regrette donc que mon amendement et ma demande d'un rapport gouvernemental ne puissent pas être examinés, mais je ne doute pas que ma proposition retiendra toute l'attention du ministère de l'intérieur,